j'informe le Sénat que de candidatures pour siéger au sein de la CMP chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelables la procédure accélérée a été engagée sur ce texte dans la discussion générale, la parole est à madame Agnès Pannier-Runacher Ministre de la Transition énergétique, vous avez la parole madame la ministre. Merci monsieur le président, madame et monsieur les présidents de commission, Madame et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, 2 tiers. 2 tiers c'est aujourd'hui la part d'énergies fossiles dans notre consommation d'énergie du pétrole, du gaz, pour l'essentiel importé du reste du monde, le nucléaire et les énergies renouvelables ne représente donc qu'un tiers de la totalité de notre consommation d'énergie. Ce qui signifie qu'à consommation égale, il faudrait multiplier par 3 notre production d'énergie bas-carbone, pour compenser la sortie des énergies fossiles. 2035. C'est la date à laquelle vingt-six de nos 58 réacteurs nucléaires arriveront au terme de 50 années d'exploitation. Tous devront alors passer le cap d'une visite de sécurité exigeante pour être prolongé, 10 années de plus. En matière énergétique 2035 c'est demain. % c'est selon RTE, la proportion d'électricité que nous devrons produire en plus à l'horizon 2050 si nous voulons enfin sortir des énergies fossiles, atteindre la neutralité carbone et répondre à nos besoins croissants. électrification pour l'industrie, les transports et les bâtiments. Mesdames et messieurs les sénateurs, ces 3 éléments montrent bien que nous sommes à un tournant historique, si nous voulons atteindre la neutralité carbone si nous voulons enfin devenir maître de notre destin énergétique, nous ne pourrons nous passer d'aucune énergies décarbonnées nucléaire comme renouvelable tant la marche à franchir est élevé, et lorsque je dis renouvelable, je veux être clair, je parle bien de toutes les énergies renouvelables, je sais que vous y êtes celles qui produisent de l'électricité mais aussi de la chaleur, géothermie, biomasse biométhane éolienne terrestre et marine hydraulique et cetera, ce que nous vivons aujourd'hui nous donne un avant-goût de ce qui nous attend demain, si nous n'agissons pas d'abord la crise climatique qui provoque les dérèglements que nous constatons tous, sécheresse, canicule feux nous vivons, nous venons de vivre en France le mois d'octobre, le plus chaud qu'on ait connu l'urgence est là, devant nous, ensuite la crise énergétique la plus grave depuis les années 70 devoir importer des énergies sans en maîtriser le coût, nous le voyons, c'est affaiblir le pouvoir d'achat des Français c'est peser sur la compétitivité de nos entreprises, c'est réduire les capacités d'action des collectivités locales face à ces enjeux, nous ne sommes pas sans solution, nous connaissons les leviers que nous devons activé pour être à la hauteur du défi, les économies d'énergie, tout d'abord grâce à la sobriété et l'efficacité énergétique, je ne reviendrai pas sur le plan sobriété que nous avons annoncé avec la Première ministre ça s'ajoute aux actions menées en matière d'efficacité énergétique, ce qu'il faut retenir c'est que d'ici 2050 nous devons réduire de 40 % notre consommation d'énergie pour atteindre la neutralité carbone la production massive d'énergie renouvelable, ensuite c'est l'enjeu du plan énergies renouvelables que j'ai lancé en juin dernier, qui a permis de débloquer 10 gigawatts de production électrique, hein térawatts de biométhane, il a aussi permis de mobiliser les services de l'État, de renforcer les équipes d'instruction sur le terrain, d'accélérer les raccordements je sais aussi que ce sont des enjeux auxquels vous êtes sensible ce texte qui vous est présenté aujourd'hui et le volet législatif de ce plan énergies renouvelables que nous allons continuer à déployer le lancement d'un ambitieux programme nucléaire, enfin, c'est la proposition du président de la République, il est désormais Soubise à une large consultation publique et afin d'anticiper, nous travaillons aussi à simplifier les procédures administratives de de construction de nouveaux réacteurs, à proximité des sites qui en accueille déjà. Tels sont les grands chapitres de notre stratégie énergétique, il nous appartient maintenant de les décliner dans une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie qui tiennent compte de la nécessité de rehausser notre ambition climatique et d'accélérer notre sortie des énergies fossiles, nous avons démarré ce travail comme nous y invite la loi en lançant en octobre une grande consultation publique, elle est inédite par son ampleur, car l'enjeu est de taille, il vous sera intégralement restituée et nourrira vos réflexions dans le cadre du projet de loi qui vous sera soumis en 2023 pour mettre à jour notre mix énergétique alors pourquoi ce projet de loi sur les énergies renouvelables, pourquoi ne pas attendre 2023. Tout simplement parce qu'à l'heure où nous voyons que nous allons devoir mettre encore plus d'ambition dans la production d'énergie, nous ne pouvons que constater que nous sommes déjà en retard sur la production des énergies renouvelables, il nous faut donc rattraper ce retard et c'est tout l'enjeu de ce projet, vous l'avez compris le combat à mener, c'est celui des énergies bas-carbone contres les énergies fossiles, c'est je pense un choix qui s'inscrit dans une position constante de notre pays depuis le cri d'alarme poussé à Johannesbourg, par le président Jacques Chirac en passant par le Grenelle de l'environnement conduit par Nicolas Sarkozy et Jean Louis Borloo ou les accords de Paris porté par François Hollande et Laurent Fabius, ce texte qui vous est présenté le fruit des échanges que j'ai eus depuis plusieurs mois avec des acteurs associatifs économiques, élus locaux et leur association et très en amont avec vous les parlementaires des différents groupes du Sénat et de l'Assemblée, à cet égard je souhaite souligner la qualité des échanges et du travail conduit par les deux rapporteurs Didier Mandelli. Et Patrick Chauvet et par les présidents des commissions du Développement durable et de l'aménagement du territoire, d'une part et des affaires économiques, d'autre part, Jean, France Longeau et Sophie Primas je tiens aussi à souligner la mobilisation de la commission des affaires culturelles et le travail qui a été menée par la rapporteure pour avis Laurence Garnier comme vous le savez je dis revoyant pas ce projet de loi à quatre objectifs, accélérer les procédures environ administrative, sans rien enlever anneaux s'exigences environnementales libérer du foncier dégradé permettre une planification par grande façade maritime pour les éoliennes marines améliorer enfin le partage de la valeur de ces projets et sécuriser le coût de l'énergie au profit des habitants, des collectivités locales et des entreprises, le texte sorti de commission montre qu'il existe en fait de fortes couvre urgence au sein des différents groupes pour aboutir à une loi qui facilite le déploiement des projets d'énergie renouvelable en remettant les collectivités au au coeur au coeur de la planification énergétique et en visant à haut niveau d'exigence en terme de nombre de projets réalisés, que ce soit l'idée d'élargir certaines mesures au biométhane, donc d'intégrer un article sur l'agro-Voltalis me, reprenant une proposition de loi largement voté sur ces bancs sur ces bancs des enrichissements été apportées et nous les soutiendrons bien volontiers la question la plus difficile reste cependant à finaliser. Celle de la manière dont l'État, les élus locaux et les porteurs de projets travaillent ensemble pour permettre un développement certes rapide, mais raisonné et équilibrée des énergies renouvelables, cela pose la question de l'implantation des projets au coeur des territoires comment répond-il aux besoins énergétiques de ces territoires, comment mobiliser associer les acteurs locaux comment minimiser autant que possible leur impact sur la biodiversité et leurs nuisances sur les communes voisines, comment ces projets se fonde-t-il dans les paysages et cohabite-t-il bien avec les habitants, au regard du retour d'expérience en la matière, certains projets sont incontestablement des succès. D'autres ne le sont pas, et nous devons le reconnaître ses échecs explique les réticences manifestes, à raison de territoire qui ne souhaite pas connaître les mêmes difficultés, cela doit nous faire réfléchir à une nouvelle méthode de conduite de ses projets, et je crois pouvoir dire au regard de mes nombreux échanges avec vous, ainsi qu'avec des élus locaux et et associations d'élus que nous sommes unanimement aligné sur ce diagnostic, ce constat d'une nécessité de changement de méthode est à l'origine de nombreux amendements que nous examinerons qui encadre plus fortement les projets d'énergies renouvelables, mais je le crains, au risque de les freiner dans ce contexte, notre responsabilité commune, hé bien de prendre en compte ces réticences tout en veillant à ne pas céder à la tentation de l'immobilisme, la question est de savoir comment notre vision de la planification énergétique n'est pas une platine fication, descendante, bien au contraire, la planification que nous appelons de nos voeux est une planification qui remet les collectivités locales et les territoires au centre des décisions je vais être très clair, le gouvernement ne reviendra pas sur la suppression de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme par le préfet, je m'y étais engagé auprès de vous, monsieur le rapporteur, ainsi qu'auprès des associations d'élus, la planification que j'appelle de mes voeux, fait des élus, des partenaires et leur donne les leviers pour agir et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté : je vous rejoins monsieur le rapporteur sur le fait que les maires doivent pouvoir avoir d'une certaine manière le dernier mot sur des projets structurants pour leur territoire, mais cela doit être précédée d'une volonté de planifier le déploiement de ces projets d'énergies renouvelables et cela peut se faire en s'appuyant sur les documents d'urbanisme nos élus peuvent davantage pour nos énergies et planifié c'est plus orientée qu'interdire accompagné nous dans le déploiement des projets nous dit ces élus car nous voulons faire, l'État doit donner le cap sur l'ensemble du pays, et être ensuite facilitateurs auprès de chaque territoire, c'est le sens de l'amendement numéro 647 du gouvernement, il propose que les élus définissent des zones prioritaires pour les énergies renouvelables, au niveau des Scott tout en maintenant les dispositions de la loi 3DS sur lesquels les sénateurs d'Arnaud et Gatel était rapporteur en permettant de prévoir des zones où le développement des éoliennes terrestres seraient encadrés afin d'inciter les porteurs de projet à déposer des projets dans ces zones, l'État pourra prévoir des bonifications dans des appels d'offres, organiser des appels d'offres dédiées à ces zones privilégiées au prioritaire de plus cet amendement donnera la possibilité au maire ou à l'EPCI de s'opposer une zone d'implantation prioritaire sur son territoire, le maire aura ainsi le dernier mot dans un processus de planification réfléchie et volontaire, au regard de cette proposition complète et équilibrée, le gouvernement demandera la suppression des articles 1er ah et 1er s'est par ailleurs s'agissant des éoliennes en mer, se pose la question des zones d'implantation de leur distance de la côte, on retrouve au fond le même type de débat en temps le ministre responsable de notre transition énergétique, je me dois de vous dire qu'à ce jour, et au regard des avancées technologiques, une distance d'implantation des éoliennes en mer, de plus de 40 kilomètres des côtes réduirait très significativement notre potentiel de développement, elle nous priverait d'un levier majeur alors qu'un parc éolien en mer de 2 gigawatts c'est l'équivalent de la production d'un réacteur nucléaire avec cette disposition, nous ne pourrons plus lancé de projet même flottant et c'est logique en mer du Nord et dans la Manche, on comprend bien pourquoi, et même en Méditerranée, compte tenu des Canyon qui existe en mer Méditerranée, seul l'océan Atlantique pourrait accueillir des projets, notamment au large de la Bretagne et des Pays de Loire c'est également je crois un très mauvais signal envoyé à des filières industrielles qui sont aujourd'hui, et c'est une chance pour la France, les plus compétitive au plan mondial, largement exportatrice, aux États-Unis, en Ecosse, elle représente près de 6600 emplois Directs, notamment à Cherbourg, au Havre ou encore hein, Saint-Nazaire, on n'a pas beaucoup de filières d'énergies renouvelables qui soient aussi puissante, prenons garde à les ménager et à les développer, c'est la raison pour laquelle le gouvernement proposera de revenir à la rédaction initiale du texte dans son amendement numéro 584 à l'article 12 au-delà de ces 2 éléments, je tiens à saluer le travail qui a été menée en commission afin d'enrichir le texte, les nombreux apports qui ont été faits concours pleinement à l'objectif d'accélération des énergies du du texte, mesdames et messieurs les sénateurs. Je suis confiante sur le fait que nous trouverons le chemin du consensus avec tous ceux et ils sont nombreux dans cet hémicycle et sur le terrain qui défendent la souveraineté énergétique et politique de notre pays. Avec tous ceux qui veulent défendre le pouvoir d'achat des Français et la compétitivité des entreprises, avec tous ceux qui veulent lutter contre le dérèglement climatique. Nous n'avons pas le luxe d'attendre pour sortir des énergies fleuve oscille, vous le savez, les Français nous regardent, je vous remercie. Merci madame la Ministre. La parole est maintenant à monsieur Didier Mandelli, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable pour dix minutes, vous avez la parole monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, une semaine après l'examen en commission, l'air, l'heure est venue d'examiner dans cet hémicycle le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelables. Je veux aussi saluer en préambule, le travail des administrateurs de la commission Vincent Carole et Victor, sans oublier Stéphanie remercier mes collègues de la commission pour leur participation aux auditions et au travail de la commission et vous remercie, Madame la Ministre, pour la qualité de nos échanges depuis plusieurs semaines, comme la commission de l'aménagement du territoire et de développement durable, la noter, c'est la première fois qu'un projet de loi est intégralement consacrée à ces énergies, c'est un signal politique fort dont nous nous réjouissons rappelons ici avec fermeté et sans ambiguïté ces énergies sont nécessaires à la préservation de notre souveraineté à l'atteinte de nos éthique de nos objectifs climatiques qu'on s'attend également avec lucidité que la France est très en retard dans leur déploiement, c'est même le seul pays de l'Union européenne de ne pas avoir atteint ses objectifs en la matière en en 2020 dans le cadre de la PPE que nous avons voté ici, nous ne pouvons évidemment nous satisfaire de ce retard qui affaiblit notre pays, notre commission par la partage donc pleinement l'objectif de ce texte : celui d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, ce constat étant dressé, nous devons, dans un second temps nous poser la question de l'adéquation de ce texte aux enjeux énergétiques et climatiques, le projet de loi qui nous a été proposé est-il suffisant, nous pouvons en douter tout d'abord, car ce texte le semble précipiter, on ne peut que regretter la méthode consistant à aborder par ce projet de loi l'exception particulier avant le cadre général, il eut été préférable, bien sûr, pour la clarté du travail parlementaire, de débattre au préalable des objectifs de développement, filière par filière, dans le cas de la loi quinquennale que nous aurons examiné en 2023 au regret, le projet de loi proposé décevant dans son ambition simplificatrice, peu de mesures du texte initial sont nature accélérer substantiellement les projets, en particulier sur le plan des procédures administratives, même en supposant que le texte proposé et son volet réglementaire lancé parallèlement cet été permettent de simplifier ponctuellement les procédures des doutes majeurs existent quant à la capacité des services déconcentrés de l'État à répondre aux besoins et instruire l'ensemble des dossiers à effectif constant, dernier grief formulé par notre commission peut déplorer de nombreux oublie et sujet non traitée dans le texte initial, fort de ces constats, notre commission souhaité relever l'ambition du texte proposé, elle a indiscutablement fait en le complétant et en l'améliorant substantiellement le premier axe de travail sur lequel nous avons avancé porte sur la planification territoriale et l'amélioration de la concertation autour des projets d'implantation d'énergies renouvelables, il s'agissait d'un véritable angle mort du texte initial, nous savons pourtant que le manque d'acceptabilité, ce qui empêche, véritablement, projets d'énergie renouvelable, de se déployer notre commission a donc proposé l'instauration d'un dispositif global de planification territoriale. Du déploiement des énergies renouvelables, je dis bien global, car l'enjeu est moins de déterminer quels documents identifierait les zones de développement des énergies renouvelables que d'instituer une méthode de concertation permettant leur identification, en cohérence avec les objectifs nationaux, nous avons donc proposé que les maires, puis les établissements publics de coopération intercommunale, en lien avec les syndicats d'énergie départements et enfin les comités régionaux de l'énergie, soit à la manoeuvre pour définir des propices à l'implantation des installations de production d'énergie renouvelable, pour ce faire, ils pourront s'appuyer sur une estimation du potentiel de production de leur territoire qui leur sera seraient transmises par l'État, une fois ces zones définies il reviendra ensuite et seulement ensuite à l'état des avalisée par décret ces zones pourront alors bénéficier de souplesse qui permettront d'accélérer substantiellement le développement des projets concernés à côté de cette planification générale, nous avons souhaité instituer une planification spatiale et temporelle spécifique au développement des projets éoliens en mer, de nombreux acteurs, critique la méthode actuelle qui consiste à développer des projets par à-coups sans visibilité quant au nombre de projets envisagés à moyen terme sur une même façade ou aux zones précis dans lesquelles ces projets pourront

afin d'orienter l'État et les porteurs de projets vers la technologie prometteuse de l'éolien flottant qui devraient arriver à maturité commerciale à l'horizon 2030 2035 j'ai également proposé que soit privilégiés, là encore, et j'insiste, des implantations de la d'une distance de 40 kilomètres du Rivage, bien entendu, il ne si j'ai pas là d'une obligation, cette règle devrait être mis en oeuvre en tenant compte des contraintes existantes sur chaque façade l'idée d'impulser une tendance à l'éloignement des parcs vis-à-vis des côtes lorsque cela est possible en laissant au gouvernement toute la latitude nécessaire autre proposition forte, nous avons souhaité renforcer la voix des élus locaux, leur permettant de s'exprimer favorablement ou défavorablement sur l'implantation d'une série de projets d'énergies renouvelables, les élus sont les plus à même de savoir quels sont les projets les plus pertinents pour leur territoire, il faut leur redonner un pouvoir décisionnaire, je l'assume car je sais que la grande majorité des élus est en faveur du développement des énergies renouvelables, faisons-leur confiance, nous avons également souhaité associer plus étroitement les particuliers, entreprises, associations et collectivités territoriales à proximité d'un site d'implantation en demandant aux porteurs de projets, de leur proposer une participation à l'investissement au capital comme cela existe au Danemark, par exemple, nous avons également largement avancé sur notre 2ème, axe de travail consacré à la simplification sur ce volet, nous allons proposer un nouvel équilibre dans la législation environnementale reposant sur 3 piliers. Le premier, plus de concertation avec le public et les élus en amont du dépôt formel des demandes d'autorisation des projets en 2, une instruction plus rapide des projets avec des dossiers de meilleure qualité, de fait, dès leur dépôt et en trois une simplification en aval pour la consultation du public avec des ajustements pragmatiques dans ce cadre, nous avons notamment proposé de supprimer certains dispositifs qui ne sont plus pertinents, à l'heure actuelle est source de charges pour les services administratifs, à l'image du certificat de projet dans le cadre de l'autorisation environnementale, nous avons souhaité également créer un référent unique au sein des préfectures de chaque département pour faciliter, instruction de tous les projets visés par le texte, tous les projets, énergies renouvelables, guichet unique référent unique et encore bien d'autres mesures, dont la création d'un fonds de garantie pour couvrir les risques contentieux, la création de nouvelles dérogations procédural temporaire. Notre 3ème axe de travail porte sur la libération de surface de déploiement à faibles enjeux environnementaux foncier, car nous sommes convaincus que notre politique de décarbonation ne nous permettra pas de relever les défis de demain si elle conduit dans le même temps au dépassement d'autres limites planétaires planétaires que sont l'érosion de la biodiversité et le changement d'utilisation des sols, nous avons donc proposé de renforcer les obligations de couverture en énergie solaire des bâtiments non résidentiels existants et nous afin d'anticiper les orientations européennes consécutives au déclenchement de la guerre en Ukraine, en contrepartie de ses obligations : nous avons souhaité faciliter l'achat de procédés de production d'énergie renouvelable afin d'équiper ses bâtiments, notamment par l'introduction d'un sur-amortissement bénéficiant aux entreprises, il nous faut également lever les contraintes réglementaires et techniques qui peuvent limiter l'installation d'ouvrages renouvelable sur les bâtiments, c'est pourquoi nous avons proposé de rendre les bâtiments neufs Solar Isablle c'est-à-dire prêts à accueillir des énergies renouvelables renouvelables en laissant la porte ouverte à toutes les innovations nombreuses par nos entreprises, nos Start-Up qui travaille sur ces sujets dans un 4ème et dernier axe, nous avons enfin souhaité sécuriser juridiquement les porteurs de projets et les autorités administratives compétentes en matière de projets d'énergies renouvelables en la matière nous ajouts sont divers et nombreux, je citerai par exemple les améliorations apportées à l'article 4 afin de garantir l'effectivité de la reconnaissance de raisons impératives d'intérêt public majeur, car en l'état du texte initial, cette reconnaissance ne pouvait concerner que les plus gros projets d'énergies renouvelables, alors que nous devons entrer dans une logique décentralisé et dans une logique d'auto-consommation en résumé ces apports de bon sens, s'appuie sur le ressort d'une plus grande achète Intelligence collective et le souci de mieux prendre en compte les réalités du terrain ou des terrains formons le voeu que le travail en séance publique nous permettent de poursuivre dans cette voie, merci de votre attention. Normaux Claire si chacun pouvait s'y tenir. Pour la suite, ce serait parfait, la parole est maintenant monsieur Patrick Chauvet, rapporteur pour avis de la commission des. Guerre économique pour cinq minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord permettez-moi parce que l'action publique n'est pas que le fait des élus, de saluer le l'excellent travail, ils se reconnaîtront d'accès d'Alexis et Coralie administrateur aux Affaires économiques, nous examinons aujourd'hui le projet de loi d'accélération de la production d'énergie renouvelables compétente en matière d'énergie et d'urbanisme, notre commission a veillé aux aspects économiques de ce texte délégation en délégation, les articles 3 16 et les titres quatre et cinq et s'est saisie pour avis des autres dispositions au cours de mes travaux, j'ai entendu 45 organismes sans personnalité et reçu 75 contributions leur constat et convergents, l'objectif du texte et partagé, mais la méthode critiquée, nous déplorons ainsi à mauvaise séquençage il aurait fallu commencer par la loi quinquennale sur l'énergie, puis examiné celle sur le nucléaire, et enfin celle sur le renouvelable. Nous regrettons aussi. Une évaluation parcellaire. On propose de modifier la facture d'énergie des Français sans étude d'un pack exhaustive. Nous dénonçons également une concertation limiter les élus locaux, comme les professionnels, nous l'ont dit, enfin, certaines mesures sont sous-calibrée, alors que la France a souscrit au plan européen visant à porter les dernières, les énergies renouvelables à 45 % d'ici 2030, rien ne garantit que cet objectif soit atteint face à la crise énergétique, nous sommes convaincus de la nécessité d'accélérer l'essor des projets d'énergie renouvelable, aux côtés de la relance de la filière nucléaire et de l'effort de sobriété énergétique pour renforcer notre transition et notre souveraineté énergétique dans ce contexte, notre commission a agi selon 3 axes : le premier axe, c'est de garantir la neutralité ne technologique entre les différentes sources d'énergies décarbonnées en comblant les angles morts du texte sur l'hydroélectricité, la commission a facilité les augmentations de puissance consolider les concessions échues ajuster les débits minimaux et simplifier les comités de suivi sur l'hydrogène, elle a intégré les conclusions de sa mission d'information sur le sujet sur le biogaz à la créer des contrats d'achat de long terme, conforter les contrats d'expérimentation simplifier les autorisations d'urbanisme faciliter les raccordements et instituer des opérations d'autoconsommation sur l'agrivoltaïsme, elle a repris in extenso la proposition sur l'agrivoltaïsme, adopté par le Sénat par 251 voix pour et 3 contre le 20 octobre dernier autre point, la commission a renforcé le critère du bilan carbone conditionnant les soutiens publics aux projets d'énergies renouvelables pour prendre en compte les métaux stratégiques et englober l'hydrogène, le 2ème axe et d'accélérer les énergies, les énergies renouvelables par l'organisation de l'État, la simplification des normes, le financement des projets et la rose, la résolution des litiges sur l'article 6 nous avons encadrer l'habilitation à légiférer par ordonnances pour qu'elle n'induise pas une érosion des compétences des collectivités, une hausse des coûts des raccordements ou une déstabilisation des rabais pour les producteurs d'énergie renouvelable et les consommateurs électro-intensifs de plus nous avons inscrit 2 dispositions en dur, la suppression d'une contribution locales et l'attribution d'une compétence à la creux sur l'article 18 nous avons ainsi réécrit le dispositif de partage territorial de la valeur pour prévoir que le reversement soient publics et collectifs et non privés et individuels, en effet, le contraire aurait été complexe à mettre en oeuvre et attentatoire au principe de péréquation tarifaire qui garantit un prix égal, de l'électricité, ce sont donc les communes et leurs groupements qui bénéficieront de ce versement, charge à eux de le redistribuer, ils devront rendre compte de son montant, et de l'allocation de plus, nous avons créé une contribution des la notation des appels d'offres, enfin, nous avons prévu que les communes et leurs groupements puissent entrer facilement au capital des sociétés dernier d'énergies renouvelables, le dernier axe et d'associer les collectivités en respectant leurs compétences et leurs finances et en décentralisant les procédures sur l'article 3 nous avons supprimé la possibilité pour l'État de modifier unilatéralement les documents d'urbanisme et au contraire fournit de nouveaux outils aux élus locaux modification simplifiée des Scott, amélioration de la planification locale articulation avec permettant d'implanter des ouvrages de raccordement en zone littorale, nous avons prévu, la vie des communes ou de leurs groupements, la priorité donnée à l'enfouissement et l'articulation avec au total nous avons infléchie et enrichi le texte en gardant toujours à l'esprit 2 impératifs, la simplification des normes crucial pour les producteurs d'énergie renouvelables et la territorialisation des projets nécessaires à leur insertion locale aujourd'hui à leur acceptation merci, allez, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à Madame Laurence Garnier, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication pour cinq minutes également. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la commission de la culture a été saisie pour avis sur le projet de loi visant à accélérer le développement des énergies renouvelables et permettez-moi à mon tour de saluer Aurore l'administratrice qui m'a accompagné dans le travail mené par la Commission au travers de notre rapport, nous avons d'abord souhaité affirmer notre conviction que la transition énergétique ne pourra se faire qu'en cherchant toujours à conjuguer et jamais à opposer développement des ENR et préservation du Patrimoine et du cadre de vie des Français, la Commission se réjouit donc des modifications apportées par la commission du développement durable pour permettre aux conseils municipaux, d'accepter ou de refuser un projet d'ENR, les maires et les élus locaux étant les premiers garants du cadre de vie des habitants, l'article 1er s'est introduit à l'initiative conjointe du rapporteur Didier Mandelli et de la commission culture nous paraît donc essentiel nous regrettons en revanche l'introduction dans le texte de dispositions qui fragilise la protection du Patrimoine, l'article onze qu'inquiet s'autorise ainsi des dérogations à l'avis conforme de l'ABF pour l'installation de panneaux photovoltaïques aux abords des monuments historiques, nous savons que les décisions des ABF peuvent parfois susciter l'incompréhension des élus locaux, toutefois cette mesure nous apparaît dangereuse pour le cadre de vie et l'attractivité touristique de nos territoires, sans apporter de gain significatif en termes d'ENR, je rappelle que l'avis conforme de l'ADF ne concerne aujourd'hui que 6 du territoire national et que même sur ces 6 pour % les avis négatifs des ABF dépasse à peine les 10 pour 100 cette mesure nous semble donc de nature à abîmer nos paysages pour un gain énergétique purement symbolique, c'est pourquoi je vous appelle à voter l'amendement de suppression que j'ai déposée. La commission vous propose également des amendements visant à adapter notre législation aux évolutions technologiques des ENR d'abord, vous le savez, la taille des a considérablement augmenté au cours de ces dernières années, les rendant désormais plus visibles sur de plus larges périmètres l'installation de nouveaux parcs et le renouvellement des parcs plus anciens plus anciens dégrade donc de plus en plus nos paysages pour prendre en compte ces évolutions, la commission présente un amendement visant à étendre l'avis conforme de l'ABF aux projets de parcs éoliens terrestres entrant dans le Champ de visibilité d'un monument historique ou d'un site patrimonial remarquable dans un rayon de 10 kilomètres et je précise qu'il ne s'agit pas d'une interdiction, mais bien dans : renforcement du contrôle afin de préserver notre Patrimoine et nos paysages dans d'autres cas, au contraire, les évolutions technologiques à l'oeuvre sont au contraire une opportunité pour préserver nos paysages et je pense à l'éolien flottant qui doit aujourd'hui nous permettre d'implanter des parcs Offshore à une plus grande distance de nos littoraux l'implantation récente du 1er parc éolien en mer au large du Croisic a suscité beaucoup d'incompréhension de la part des élus locaux, soucieuse de préserver nos littoraux de l'impact visuel et de l'effet d'encerclement que j'ai moi-même constaté dans mon département de la Loire-Atlantique, la commission vous invitera donc à interdire l'implantation de ces parcs à moins de 40 kilomètres des côtes à compter des prochains appels d'offres. Personne ici ne conteste le développement des ENR et leur nécessité pour faire face aux enjeux d'écologie et de souveraineté énergétique mais veillons aussi à ce que leur déploiement ne constitue pas un nouveau motif de fractures et de divisions sociales et territoriales. Alors que les éoliennes terrestres se développe aujourd'hui souvent en milieu rural et souvent en milieu rural, pauvre, une étude qui date de 2019 a montré que les manifestants pour le climat était majoritairement jeunes urbains et issus de classes sociales privilégiées, si l'on veut, mes chers collègues, que les enjeux écologiques ne soit pas porter uniquement par quelques-uns, mais bien partagée par tous les Français nous devons tracer cette ligne de crête et trouver le bon équilibre entre ENR et cadre de vie, reprenons : discours de Malraux qui défendait sa loi en 1962 et qui imaginer des quais de Seine, livré sans règle au promoteur. Malraux disait si nous laissions détruire ces vieux qui est de la scène semblable à des lithographies romantique, il semblerait que nous fassions le génie de Daumier et l'ombre de Baudelaire, n'oublions pas que nos prédécesseurs ont su préserver et protéger ce Patrimoine français qui a fait de notre pays, la première destination mondiale, notre responsabilité est donc bien aujourd'hui de conjuguer développement des énergies renouvelables, avec les enjeux économiques et touristiques territoriaux et sociaux pour que notre pays soit au rendez-vous de toutes ses ambitions.

Merci monsieur le président. permettez-moi d'abord de remercier mon collègue Didier Mandelli, non seulement pour le travail effectué, mais aussi pour avoir ouvert l'ensemble de ces auditions à tous les collègues qui le souhaiter, mes chers collègues, il y a très exactement une semaine nous débattions de la politique, j'ai énergétique de l'État pour le présent projet de loi constitue l'une des déclinaisons opérationnelles si José la métaphore culinaire, je dirais que dans le menu qui nous a proposé le chef de l'État lors de son discours de Belfort, le projet de loi initial, telle que nous est soumis, apparaît comme une recette bien alléger et qui manque cruellement d'ingrédients le sujet aurait mérité une approche globale et je suis convaincu qu'un temps de maturation plus long aurait permis d'aboutir à un texte plus cohérent, intégrant l'ensemble des énergies renouvelables, je pense à l'hydrogène à l'hydroélectricité cher à Monsieur Grimm, mon collègue Gremillet au gaz vers l'agrivoltaïsme, ou encore l'énergie marémotrice sur l'agrivoltaïsme nous comprenons mal dans notre groupe que l'amendement de notre collègue Nathalie Delattre proposant d'intégrer les fermes pédagogiques au dispositif était déclarée irrecevable de l'Arctique 40, franchement, mes chers collègues, refuser un investissement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments d'établissements scolaires agricoles qui non seulement produit l'énergie, mais aussi de surcroît pédagogique pour ses futurs jeunes agriculteurs brandir l'Arctique quarante c'était vraiment abusé le travail de ne de commission à Foro heureusement pu enrichir le texte et je me félicite, en particulier des avancées concernant l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, nous aurons à débattre encore et je sais que nombre de nos collègues ont déposé des amendements sur cette question globalité aussi dans l'approche de la question énergétique elle même alléger les contraintes administratives pour accélérer les projets est une chose mais qu'il nous faut aussi créer les conditions pour réussir cette transition, l'adaptation des réseaux qui doivent devenir intelligents, organisation du stockage de l'énergie produite, qui est un vrai défi, la structuration d'une véritable filière industrielle, la nécessaire recherche en parallèle d'une réduction de nos consommations par l'automatisation des outils de pilotage et surtout de nos comportements, la décarbonation de notre économie qui repose, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, encore dans notre pays, à plus de 60 % sur les énergies fossiles, nous ne pouvons faire l'économie de ces sujets urgents,

je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur les motifs mis en avant, en particulier sur la question de la lenteur des procédures, c'est un procès récurrent fait à nous, administration, mais la principale cause d'anciens a-t-il pas le manque de ses moyens humains et financiers, nous vivons dans tout son quotidien dans nos territoires, l'État depuis longtemps s'est désengagé, les effectifs des directions départementales ont fondu comme neige au soleil, nos services déconcentrés, ce sont bien souvent en panne sèche, mais Madame la Ministre, on nous avait heureusement rassuré sur cette thématique dans le même temps, le texte doit restaurer la légitime place des collectivités, elles sont aux côtés des habitants, les premières concernées par les impacts des nouvelles installations, comme l'a dit très justement Madame la Ministre, en charge des collectivités, interrogé sur les ânes, elles sont les mieux placés pour évaluer leurs besoins, leurs contraintes et pour chaque dispositif sur les principes d'adaptation de planification de programmation de territorialisation qui doivent s'imposer là aussi notre commission a d'ores et déjà améliorer le texte, il ne faut aller plus loin, aussi je salue les dispositions du projet de loi qui vise à créer un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables ou imposer aux sociétés de projets de proposer des parts aux résidents et aux collectivités, cependant, la très grande majorité de mon groupe s'opposera au droit de véto des collègues quitté sur les projets d'installation d'éolien terrestre du biogaz ou du photovoltaïque, ainsi qu'à la distance minimale des 40 kilomètres des côtes en matière d'éolien en mer, de manière générale, parce que les enjeux pour les générations futures sont colossaux, nous devons ça Jean de la question de la simplification des procédures, faire preuve de responsabilité, de lucidité, trouver le juste équilibre entre la préservation de notre environnement et la nécessité d'accélérer notre transition énergétique sans céder à l'arbitraire ni oppression de ce point de vue, je reste convaincu, plus que jamais que les principes de proportionnalité et de réalisme doivent nous guider, je prendrai un seul exemple désolé, celui de l'amendement relatif à la suppression de l'avis conforme des ABF pour l'installation de panneaux solaires sur les toits des habitations en proximité de sites classés une avancée bienvenue, sachons préserver notre Patrimoine mais soyons aussi raisonnable, vous verrez qu'on pris mes chers collègues, notre groupe adoptera une attitude très constructive sur ce texte, tout en restant attentif aux impératifs de démocratie participative et aux enjeux de la préservation de richesses naturelles, je vous remercie. Merci. Collègue, la parole est maintenant à ma Madame Marta de Cidrac pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre Mesdames Madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, nos concitoyens regarde avec inquiétude leurs factures d'énergie, il se questionne et s'inquiète car autour de nous en Europe, les compteurs s'affolent, l'électricité est en hausse de 80 % au Royaume-Uni 55 ans en Belgique 45 aux Pays-Bas, une seule réponse : produire plus une électricité abondante disponible et bon marché, voilà la réponse que les Français attendent, à défaut d'être la réponse attendue ce texte a le mérite d'être une réponse les vertus environnementales du renouvelable ne sont plus à démontrer, et est de la France à tenir ses engagements internationaux en matière d'émission je salue la volonté du gouvernement d'amplifier notre production d'énergie bas-carbone Il était temps, c'est un chemin qui, je l'espère, augure aura d'autre déclic à regret malgré tout celui d'une politique énergétique subie et non choisie au coup par coup, un jour, on fragilise le nucléaire, le lendemain on promeut les ENR demain en réhabilitant le nucléaire, un autre jour, on saluera l'hydrogène, tout cela est brouillon et manque de cap et de vision, nous aurions certainement gagné à avoir un grand débat sur la stratégie et l'avenir énergétique de la France, cette volonté d'amplifier, de diversifier notre production bas-carbone n'émerge pas de nulle part, comme ailleurs dans le monde, nous sommes rattrapés par la réalité d'un dérèglement climatique incontestable et d'un contexte international dégradé qui vient bousculer des approvisionnements et des échanges commerciaux que nous croyons pérenne, mais la réalité internationale ne doit pas nous faire oublier la réalité nationale, là même qui depuis 10 ans à contribuer à affaiblir notre production énergétiques bas-carbone et à fragiliser l'autonomie énergétique de notre pays, accélérer les ENR demain oui pour faire oublier qu'hier on a fermé Fessenheim renoncer au projet Astride, vendu, puis racheté à Alstom Power repousser le grand carnage ou encore échoué à pérenniser les EPR qu'avons-nous fait de notre indépendance énergétique qui garantissait à la France une énergie abondante disponible et bon marché, aujourd'hui, c'est sur le charbon que nous comptons pour compenser nos réacteurs arrêtés et sur le gaz que nos concitoyens compte pour espérer se chauffer, alors évidemment, faisons en sorte que demain nous puissions pleinement compter sur le secteur du renouvelable dans le mix énergétique français mais Madame la Ministre, combien de kilomètres carrés de Champ photovoltaïque, combien de kilomètres de côtes garni d'éoliennes en mer, faudra-t-il pour répondre aux besoins de la France et quelles précautions devront nous prendre en matière environnementale et de souveraineté énergétique telle doit être la contribution de ce texte aux grands enjeux énergétiques de demain, telle est son ambition et je l'approuve, pourtant il élude certains sujets essentiels, accélérer la production des ENR signifie leur déploiement massif partout dans les territoires, s'interroger sur leur impact environnemental et économique et salutaire est crucial, soyons lucides, les déployer sans discernement ni quelques précautions signifierait financer une industrie venus d'ailleurs constat regrettable mais que chacun connaît les géants industriels de cette filière sont aujourd'hui principalement chinois pour le photovoltaïque danois et allemands pour l'éolien et l'éolien en mer je souhaite en effet que les entreprises français se saisissent de ces opportunités environnemental, économique que le texte laisse entrevoir et veillons, madame la ministre, à ce que dans les différents plans d'investissements d'avenir et plan France 2030, nous encourageons les initiatives françaises et que nous les soutenions ne réitérons pas les erreurs du passé, nous n'avons pas su créer une filière industrielle française d'équipements compétitifs et vertueux sur tout leur cycle de vie, les traitements des déchets et le recyclage sont également un enjeu impératif des équipements démantelé accélérer aujourd'hui les implantations c'est demain devoir en subir le coût environnemental avec tout ce que cela comporte en terme de traitement et de valorisation des déchets pour le photovoltaïque, une filière REP s'est structuré, ce qui n'est pas à ce jour le cas pour l'éolien, l'échéance et pourtant déjà là car d'ici 2025 les premières générations d'éoliennes devront être démantelées selon l'Ademe, la masse d'une éolienne et recyclables à 90 % l'essentiel de la masse et dans ses fondations et des filières existent en effet pour les fondations, mais ce n'est pas le cas pour tous les composants, comme les pales, par exemple, or si nous accélérons le déploiement des éoliennes, il est impératif d'anticiper le traitement de tous les déchets issus de leur démantèlement anticipons dès maintenant, ayons une vision d'avenir à 30 ans sur l'ensemble du cycle de vie des éoliennes implantées dans un souci d'économie circulaire, je me réjouis de l'adoption en commission de mon amendement visant à créer une filière REP ou tout système équivalent de prévention et de gestion des déchets pour l'éolien, avant de conclure : je souhaite aussi remercier notre rapporteur Didier Mandelli pour son écoute tout au long de l'examen du texte et pour tout le travail effectué au sein de notre commission ce texte enrichi par l'apport de tous les commissaires va sans mauvais jeu de mot de ma part, libéré des énergies pour un secteur qui ne demande qu'à se développer, mais pour que le déploiement sont ambitieux, accepté dans nos territoires, Madame la Ministre, il faudra tenir compte de l'ensemble des enjeux importants. Madame de Cidrac je vous remercie. Merci à chacun de respecter les temps je rappelle que. Il y a 573 amendement si chacun déborde, moi ça m'est égal, je préside samedi après-midi mais bon. Allez la parole et il a bien fait de monter toute de suite à monsieur Pierre vielle pour les indépendants pour cinq minutes. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, la guerre en Ukraine et ses conséquences géopolitiques et économiques en bouleverser les circuits d'approvisionnement des produits énergétiques fossiles rappelant la dépendance de notre économie et de nos modes de vie aux énergies importées, cette situation constitue un nouveau paradigme, donc il nous faut prendre acte dans ce contexte, le gouvernement a présenté ce projet de loi ayant vocation à répondre rapidement et efficacement aux défis énergétiques que nous aurons à relever dans les années à venir, c'est un signal politique fort, je tiens d'abord à saluer l'oreille très attentive du gouvernement dans la phase de préparation de ce texte, mais aussi le travail effectué au sein de chaque commission qui a notamment permis l'adoption de plusieurs amendements déposés par des sénateurs de notre groupe sur des points essentiels. Vous le savez, le groupe les zen de pendant soutien une écologie libérale pragmatique et pertinentes à l'nous devons absolument aller vers une simplification en matière de déploiement de dispositif générateur d'énergie renouvelable ici simplifier implique de réduire le temps de développement d'énergie renouvelable pour accélérer leur déploiement sur nos territoires simplifier inclut également de libérer des énergies et des technologies nouvelles pour gagner, en souveraineté, notamment grâce à la production de nerfs et bas carbone ces dernières constitue selon moi une Pierre angulaire de notre mix énergétique qui à terme dont nous permettre d'assurer notre alimentation en électricité tout en préservant notre environnement. Par ailleurs, si le projet de loi actuelle couvre un large spectre de solutions énergétiques, il a dû être complétée afin d'y inclure l'hydrogène la géothermie ou l'agrivoltaïsme. En effet, il me semble essentiel que l'agrivoltaïsme puisse figurer dans ce texte au sein de sa niche parlementaire du 20 octobre dernier. Le groupe, les indépendants a porté et fait adopter une proposition de loi visant à encadrer le développement de ce pratique. Ces mesures ont pu être inséré dans le texte dès l'examen en commission, j'en profite pour remercier les auteurs des différents amendements déposés, l'agrivoltaïsme n'importe tout particulièrement puisque, rappelons-le, ces bénéfices sont multiples, il permet à nos agriculteurs d'avoir un revenu complémentaire tout en garantissant la primauté de l'activité agricole. Il représente également une nouvelle source de production énergétique sans aggraver l'artificialisation des sols, point essentiel qui est revenu dans mon débat certes je viens d'évoquer des avancées tout à fait notable pour autant le travail doit se poursuivre, je suis convaincu que nous devons penser leur transition dans une architecture plus large, c'est pourquoi les autres textes annoncés. Dès le début de l'année prochaine, me semble indispensable afin de poursuivre nos objectifs vers davantage d'indépendance énergétique. Parmi ces textes, je pense à la programmation pluriannuelle de l'énergie ou encore au projet de loi sur le nucléaire, énergie qui restera essentielle dans notre mix et énergétique décarboné. Rappelons également l'importance du stockage des ENR question absente jusqu'ici, le stockage de ces énergies dites intermittente présente un potentiel important, notamment grâce à la technique du power to Go qui, pour le dire plus simplement tient à transformer les ENR en hydrogène. Une dernière problématique me tient à coeur, il s'agit de la place des collectivités locales et des élus locaux dans le développement des ENR, je suis convaincu du rôle qu'ils ont à jouer en la matière, mais je crois aussi en l'importance de trouver un équilibre juste entre un droit de véto qui leur seraient octroyés pour l'installation de projets ENR et l'impératif de développement des énergies renouvelables et bas carbone, la question peut paraître clivante mais nos besoins énergétiques immédiats sont une réalité et ne peuvent souffrir d'un droit de blocage qui seraient souvent arbitraire. De même, je ne suis pas du tout persuadé que l'octroi des autorisations en matière de dispositifs d'énergies renouvelables au seul maire serait le rendent service il se retrouver dans tous les cas, seul sous une autre forte pression, voir le communiqué national de l'AMRF à travers ce texte nous devons privilégier le sens de l'intérêt collectif et mettre de côté les intérêts politiques partisans. En matière d'énergies renouvelables, le meilleur reste à venir, je pense, je pense par exemple au projet d'Airbus Defence and Space toulousain sur leur bim centrale photovoltaïque spatiale. Qui pourra alimenter les avions en vol par faisceau notre indépendance énergétique dépendra également de notre audace de notre ambition et des futurs progrès technologiques notre gros pour les indépendants votera en faveur de ce projet de loi pour soutenir l'effort commun vers une transition durable et vers davantage de souveraineté énergétique. Merci, cher collègue, la parole est maintenant monsieur Ronan Dantec, pour le groupe écologiste pour cinq minutes. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs et Madame, les rapporteurs, monsieur le président de commission, chers collègues, enfin, enfin, l'État reconnaît que face à la très grave crise énergétique que nous vivons, nous n'avons qu'une seule solution : le développement rapide et massif des énergies renouvelables, notamment pour la production d'électricité, les seules loi arrive malheureusement bien tard presque 8 ans après que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte est déjà fixé à l'horizon 2025 le rééquilibrage du mix énergétique français entre le nucléaire et les énergies renouvelables c'est un temps suffisant pour développer une réelle stratégie territoriale et industriel mettre en cohérence dans les politiques publiques, les objectifs fixés par la loi, mais force est de constater que ce temps a été gaspillé pour des raisons que je n'aurait guère le temps de développer et au détriment, donc de notre économie et du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, nous sommes aujourd'hui le seul pays européen à ne pas tenir les objectifs de développement des énergies renouvelables, prévue dans la directive cadre de 2009 en urgence, donc le gouvernement nous dit son intérêt son empressement pour les énergies renouvelables que Madame la Ministre a qualifié hier matin sur une grande radio nationale, je la cite d'ultra-compétitif rejoint donc par l'État dans l'analyse que notre salut passe par les énergies renouvelables, une question de survie, a aussi dit madame la première ministre le groupe écologiste solidarité territoire accueil donc évidemment favorablement cette loi mais car il y a un mais, s'interroge quand même un peu sur son efficience 1er point le retard du développement des énergies renouvelables et d'abord actuellement lié au prix trop bas proposés par la Commission de régulation de l'énergie, la creux qui ne permettent pas le succès complet des appels d'offres si clairement les énergies renouvelables produisent aujourd'hui l'électricité la moins chère et tarifs proposés sont néanmoins trop bas, j'entends bien sûr, Madame la Ministre votre préoccupation de ne pas créer de super-profits injustifiés pour les entreprises du secteur, surtout vous vous interdis rien en plus de l'Hérault taxé après mais même avec quelques euros de plus sur ce prix, les énergies renouvelables resteront de loin les moins chers, ensuite, la deuxième raison du retard est lié à la prudence des investisseurs qui attendent que tous les recours, même les non suspensif soit expurgé sur ce point, l'amendement du rapport de la commission du rapporteur de la commission du développement durable, dont je salue moi aussi l'engagement sur ce texte, a très opportunément ouvert à la création d'un fonds de garantie mutualisant les risques liés au recours contentieux, c'est probablement le dispositif qui nous permettra de gagner le plus de temps dans la mise en oeuvre des projets ainsi les gains espérés sur les simplifications administratives qui sont le socle du texte apparaissent assez secondaire par rapport au point que je viens d'évoquer le groupe écologiste est très vigilant sur le fait que ce texte ne détricote pas le droit de l'environnement et ne s'applique pas en dehors du sujet des énergies renouvelables et n'affaiblisse donc pas le la non-régression du droit de l'environnement, le gouvernement a entendu l'avis très négatifs et ferme du Conseil national de la transition écologique et le texte a été modifiée dans le bon sens depuis sa première présentation certains points reste néanmoins problématique, notamment sur les enjeux de biodiversité, nous y reviendrons durant le débat en séance, reste les lignes rouges allègrement franchi par la majorité sénatoriale qui a fait de ce projet de loi, un texte de ralentissement plus que d'accélération, le droit de véto des maires pour des projets qualifiés par ailleurs comme relevant de l'intérêt général est assez étonnant, voire même de l'ordre de l'oxymore, c'est d'ailleurs un revirement historique de la part d'un mouvement aux racines gaullistes et jacobine toujours fier de mettre en avant les épopées industrielles du pompidolien isme et si c'est donc l'inverse, l'intérêt national s'face face aux enjeux locaux, c'est une première qui ouvrira demain à la porte à l'un titre édition par décision locale ici d'un bout de ligne de TGV et pourquoi. Pas là-bas, d'un petit réacteur nucléaire, ça va devenir très complet, alors voilà une stratégie nationale de même. Plus vous l'interrompez plus je vais lui donner du temps de parole alors bon c'est pas le faire. faire. Allez, allez, on se calme, ce mal. ça va donc devenir très compliqué d'avoir une stratégie nationale de même renvoyé à 40 kilomètres les éoliennes en mer, on interdit le développement sur la majorité du littoral, je veux bien qu'un léger inconfort pour des propriétaires de résidences secondaires, avec vue sur mer soit plus important que l'a dit, l'avenir de notre industrie et la facture énergétique des Français et Françaises mais je m'interroge quand même sur le sens de certaines priorités le maintien de ces de barrière va rendre évidemment ce texte nos tables en l'état pour le groupe écologiste, mais nous espérons néanmoins que le bon sens collectif l'emportera durant les débats en séance. Merci et. La parole est maintenant madame Nadège avait pour le groupe RDPI pour six minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, monsieur le rapporteur Mandelli madame la rapporteure, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, notre maison brûle et nous l'avons vu concrètement cet été avec 66000 hectares partis en fumée en Gironde, dans les Landes et même dans le Finistère, le mois d'octobre, c'est qui s'est achevée, aura été le plus chaud de notre histoire, face à cette réalité à cette menace d'un réchauffement climatique de près de 3 degrés l'ONU il y il y a quelques jours, rappelait que l'unique option était la transformation rapide, urgente de nos sociétés à l'occasion du lancement du Conseil national de refondation Climat et biodiversité la première ministre a également alerté sur la radicalité des changements à effectuer afin de franchir la marche avec cet objectif d'atteindre la neutralité carbone en milieu de siècles le défi à relever est colossal et la fenêtre d'opportunité est en train de se refermer à plus court terme, face à des circuits d'approvisionnement en pétrole et gaz mis à mal par la guerre en Ukraine, il est aussi nécessaire d'activer tous les leviers, il nous faut en effet développer toutes les sources d'énergies décarbonnées notamment renouvelable, en particulier l'éolien, le photovoltaïque ou encore la méthanisation il nous faut accélérer une nécessité, alors que notre pays, il est vrai, est en retard en 2020 la part de ces énergies dans la consommation finale brute et d'environ 19 % 3 points de moins que la moyenne dans l'Union européenne sur la base de ce constat, ce texte constitue une réponse à laquelle il faut ajouter, bien entendu, l'entretien et le développement de notre parc nucléaire pour défendre notre souveraineté maîtriser les coûts et atteindre la neutralité carbone il y a une semaine, notre commission a adopté 129 amendements et je veux ici saluer l'engagement sur ce texte de notre rapporteur Didier Mandelli qui nous a permis d'assister aux auditions ainsi que celle de la ministre, Madame la Ministre, pour votre écoute le titre hein, du projet de loi entend apporter des mesures d'urgence notamment procédurale pour accélérer les projets d'énergies renouvelables et industriels, notre commission a pu ajouter, préciser des dispositions utiles à ses premiers articles, je pense notamment à la désignation des référents préfectoraux dans chaque département pour l'instruction des autorisations relatives au projet de ENR d'autres modifications ne nous conviennent pas, et j'y reviendrai, afin d'accélérer le développement de l'énergie solaire, qui est l'objet du titre suivant le texte auront notamment possible l'installation de ses ouvrages

mais adaptée aux enjeux contemporains, c'est dans cette logique que je soutiendrai en séance plusieurs amendements déposés sur l'article 9, nous avons également fait adopter en commission de dérogation, sur le modèle des antennes relais dans la loi et long. Afin que soit demander un avis simple de l'architecte des Bâtiments de France pour un projet d'installation à des fins d'autoconsommation sur les bâtiments situés en zone classée avec des conditions précisées par décret, je m'en expliquerai lors des échanges à venir, mais j'ai eu de très bons retours des élus de mon territoire sur cette proposition, il s'agit de la même philosophie pour l'agrivoltaïsme, qui constitue une grande réserve de foncier, si la pas très pratique, est faite de manière régulée, sans mettre en cause l'activité agricole. à ce propos, mon groupe tient à remercier nos collègues pour leur travail qui a abouti à une proposition de loi équilibrée et raisonnée, adopté il y a 2 semaines, dont les dispositions ont été introduites dans le texte sur le développement d'éolien en mer ensuite dans le pacte signé il y a quelques mois, l'État a confirmé sa volonté d'un déploiement ambitieux avec un objectif d'attribution de 40 gigawatts d'ici 2050, la filière s'est engagé quant à elle a quadruplé le nombre d'emplois Directs et indirects liés à l'éolien en mer d'ici 2035 et engagé plus de 40 milliards d'euros d'investissements en 15 ans. Une filière structurée, donc en forte croissance mais qui a besoin de visibilité de planification et nous aurons l'occasion d'y revenir pendant les débats, c'est une filière qui a aussi besoin d'être conforté, aussi nous voterons contre le seuil des 40 kilomètres cela reviendrait sur la Côte d'Opale à ne pouvoir en faire du tout ou alors sur le territoire britannique, plus sérieusement une telle distance au large de nos littoraux serait contraire à une planification territoriale équilibrée de cette énergie aussi sur l'éolien terrestre, nous avions trouvé un juste équilibre à l'issue de l'examen de la loi 3DS or, ce qui a été votée en commission revient à donner un coup d'arrêt au projet de construction des d'exploitation que des concertations locales et lieu évidemment et nous soutenons que les les élus locaux puissent intervenir sur des projets d'implantation dans le cadre d'un échange encadré avec le porteur de projet, mais nous sommes opposés au droit de véto. Telle que définie, position partagée notamment par l'Association des maires de de France dans leur communiqué de presse du 2 novembre parmi les deux les dispositions relatives au financement et au partage de la valeur, il nous est apparu nécessaire de soutenir des mesures d'appropriation et des modèles de financement locaux. Au service des territoires, c'est pourquoi nous avons déposé un environnement qui a fait objet de faciliter le développement de l'auto-consommation de gaz renouvelable, c'est dans ce même esprit d'efficacité et de diversification que nous avons déposé un amendement de séance pour que les acheteurs publics puisse recouvrir en toute sécurité juridique aux nouveaux modes de commercialisation de l'électricité d'origine renouvelable que sont l'autoconsommation, les contrats d'achat délicat. Renouvelable, ce sont des mesures facilitent gestatrice mais Simple qui pourront s'avérer très utile pour nos collectivités et nos PME, en conclusion, notre groupe suivra toute proposition toutes les idées qui peuvent soutenir et renforcer le développement des énergies décarbonnées et à contre-travail nous nous opposerons à toutes celles défensives qui un truc qui ils traduiront par une décélération, je vous remercie.

Monsieur le président, madame la ministre, Madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, tout le monde s'accorde à dire que nous devons accélérer le développement des énergies renouvelables, en particulier pour faire face à la demande croissante en électricité qui viendra se substituer, notamment dans les transports et l'industrie aux énergies fossiles, rappelons tout de même que notre production actuelle d'électricité grâce à son mix énergétique et faiblement carbonée, la crise énergétique les lié à l'agression de l'Ukraine par la Russie nous fait mesurer combien il est urgent d'agir, et peut être regretter que les grandes orientations stratégiques et la planification qui en découle n'ait pas été anticipé au cours du précédent quinquennat ce projet de loi est certes le bienvenu, mais il aurait été plus logique de procéder de façon rationnelle en élaborant de façon concertée, la stratégie française pour l'énergie et le climat une stratégie globale comprenant certes la production mais aussi la sobriété, l'efficacité énergétique avec l'intensification des procédés industriels, mais aussi l'isolation thermique des bâtiments et puis enfin la captation par les pluies carbone tout cela nous est annoncée pour 2023 avec une loi de programmation pour l'énergie et le climat, ainsi qu'une 3ème PPE qui couvrira les périodes 2024 2033 ainsi aussi qu'une 3ème stratégie nationale bas-carbone et enfin un plan national d'adaptation au changement climatique, alors dans ce contexte, nous devons analyser ce projet de loi avec pragmatisme, en essayant d'anticiper tout ce qui peut l'être et en posant des accroches qui pourront servir d'appui à la future stratégie en ayant pour boussole le principe que l'accélération ne doit pas se faire ni au détriment de la concertation, ni au détriment de l'environnement, la concertation et les procédures qui en découlent sont souvent perçus comme un boulet qui freine les projets alors qu'au contraire la concertation en amont, plus elle associe la population et les élus plus alors les projets sont faciliter la concertation fluidifie les procédures son absence, les crises et les le le rapport du Conseil économique, social et environnemental acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique transition subit transition est éloquent dans ce domaine, le texte qui nous est soumis, a été profondément remodelé par les commissions sénatoriales et je dois moi aussi souligner l'implication des rapporteurs et cette réécriture comporte de nombreuses avancées avec l'introduction d'une planification territoriale, même si l'on doit se poser la question de l'échelle pertinente et de la méthode, la mise en place d'une concertation préalable systématique la désignation d'un référent départemental préfigurant un guichet unique mais qui renvoie, aux moyens dont l'État dispose pour instruire et accompagner les projets la création d'un fonds de garantie l'extension à de nombreux bâtiments de l'intégration d'un procédé de production d'énergie renouvelable, sur une surface de leur toiture, la prévention des par des pratiques de dumping social sur les navires dans les parcs éoliens en mer, la création d'un mécanisme de suramortissement et enfin la mise en place d'un nouveau dispositif de partage de la valeur, mais hélas ce qui a été accordé d'une main pour faciliter les projets semblent avoir été repris de l'autre, en ajoutant des verrous qui vont compliquer les déploiements la majorité sénatoriale, MU, sans doute par un tropisme vendéen risque de transformer la vie des porteurs de projets en épreuve de Fort Boyard, le rejet implicite le rejet implicite de l'éolien en mer au-delà des 40 kilomètres condamne l'éolien imposé en Méditerranée, il exclut la quasi-totalité de la mer de la Manche et de la mer du Nord et fragilise de sorte la filière industrielle française qui s'est implantée en créant des emplois sur Le Havre, Cherbourg et même Saint-Nazaire car la technologie française de l'éolien flottant n'est pas encore arrivé à une totale maturité dans un autre domaine, même si l'on comprend et partage l'exaspération des élus locaux, à qui l'on a quasiment imposer des champs d'éolien terrestre, il est légitime de se poser la question s'il n'y a pas des moyens consensuels, basée sur l'Intelligence collective des territoires pour trouver des solutions et substituer à la décision individuelle, une décision collégiale, je ne doute pas que ces sujets animeront nos débats et c'est en fonction de ce texte définitif et les amendements adoptés que le groupe ce que notre groupe déterminera sa position. Merci, cher collègue. La parole est maintenant Madame Marie-Claude va Ayaz pour le groupe CRCE pour cinq minutes. Merci monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur dans son dernier rapport, le GIEC alerte sur la nécessité de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et pour cela identifie des solutions possibles dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'industrie et de l'usage des Terres, il insiste néanmoins sur la nécessité d'une transition juste tant les inégalités sont flagrantes au niveau mondial les 10 pour 100 des plus riches sont à l'origine de 36 à 45 % des émissions quand les pays les plus pauvres ne sont responsables que de 3 à 5 en matière de déploiement des ENR nous faisons figure de mauvais élève puisque nous sommes le seul pays à ne pas avoir atteint notre objectif de 23 % dans notre consommation finale d'énergie lorsque l'on sait que l'objectif est de 33 % à l'horizon 2033 si le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste est favorable au développement des énergies renouvelables au côté de notre mix énergétique historique d'origine nucléaire et hydraulique nous considérons cependant qu'elles ne doivent pas être génératrice de nouvelles dérégulations et que leur essor exige la structuration de véritables filières par la puissance publique, nous savons que la théorie qui consiste à laisser faire le marché s'avère extrêmement coûteuse pour les usagers, ce projet de loi en défendant une accélération intensive des projets plutôt qu'une planification réfléchi en amont propose la manière forte avec le risque de s'avérer contre-productive en radicalisant les oppositions et en éloignant les citoyens des enjeux de la transition énergétique à l'occasion de la concertation que vous n'avez pas manqué, Madame la Ministre d'organisé autour de ce texte, nous n'avons pas manquer aussi non de vous renvoyer la voix de nos territoires, élus, associations, citoyens qui, face à des implantations quasi imposé exigent légitimement de prendre toute leur place en amont des projets, le rapport présenté au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable par notre collègue rapporteur Didier Mandelli qui remanie, ce projet de loi de 129 amendements, insiste sur les avancées nécessaires en matière d'accepter dès que ça d'acceptabilité et de planification des projets mais il demeure cependant dans ce texte des adaptations de procédures administratives qui constituent des reculs démocratiques comme notamment la consultation des citoyens par la voie électronique alors que ce sont précisément les territoires concernés par ces implantations qui sont les plus éloignés du numérique à cet égard, d'ailleurs, je cite le Conseil économique, social et environnemental, qui recommande d'aller chercher la contribution des personnes silencieuse et des invisibles, en veillant à prendre en compte l'électronique, il prône aussi d'ailleurs aussi l'évaluation a posteriori de la concrétisation des engagements des porteurs de projets, la procédure simplifiée de modification des documents d'urbanisme et de nature, elle aussi à faciliter les atteintes à l'environnement par ailleurs et vous le savez madame la Ministre, ces nouvelles procédures accélérées ne pourront être efficiente ça renforcer les moyens humains, des services de l'État, comme ne manque pas d'ailleurs de le relever, le Conseil d'État, ce projet de loi défend un modèle visant à décor décarboner la production qui sont doit aller de Pair avec la notion de sobriété, vu sous l'angle par exemple du soutien aux transports collectifs dans le ferroviaire et l'isolation thermique des bâtiments face au prix de l'énergie face aux attentes des Françaises et les Français, nous devons être le plus efficace possible 13 millions de familles vivent aujourd'hui dans ce que l'on appelle des passoires thermiques et qui souffrent, qui souvent se chauffe dans des conditions déplorables, comme nous le rappelle les 3000 intoxications au monoxyde de carbone qui ont lieu chaque année, il y a urgence à soutenir un grand plan de lutte contre la précarité énergétique en capacité de créer des emplois non délocalisables, avec de vrais résultats en terme de confort et de pouvoir d'achat des ménages par ailleurs mon groupe ne soutiendra pas les modèles de financement hybride promu dans ce texte, en matière de partage de la valeur ce système aboutit à différencier le prix de l'énergie en fonction de la localisation des clients et en compte, contrevenant ainsi gravement au principe d'égalité entre les usagers s'il doit y avoir un retour économique liée à la présence de ces installations, alors il doit revenir aux collectivités locales qu'hier j'qui elle gère l'intérêt général, l'énergie est un bien commun, un droit fondamental et universel car il permet l'accès au droit aux autres droits que sur le lot, l'accès à l'eau à la santé, à l'éducation à l'emploi à l'insécurité à l'égalité entre les hommes et les femmes, la libéralisation des marchés de l'électricité, engagé en 1996 a conduit les à l'éclatement du service public de l'électricité et du gaz, les ENR doivent être sorti des griffes du marché pour être développés là où elles sont le plus efficace en ayant pour critère l'intérêt collectif et celui de la protection de l'environnement si effectivement ce projet de loi amendée par la commission comporte quelques avancées notre vote dépendra des débats et des amendes de qui en résulteront, je vous remercie. La parole est maintenant madame Denise Saint-Pé pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le texte que nous allons examiner aujourd'hui revêt une importance toute particulière alors que nous connaissons une crise énergétique sans précédent à l'heure où le spectre d'une pénurie d'énergie resurgit d'autant plus menaçant que notre parc nucléaire et pour moitié indisponible, il est en effet plus nécessaire que jamais d'accélérer notre production d'énergie renouvelable, cela permettrait d'éviter Rano ménages nos entreprises et nos collectivités locales de subir délestage rationnement ou black-out, tout en garantissant notre souveraineté énergétique et en s'inscrivant dans la lutte contre le changement climatique, il ne s'agit pas pour autant de négliger le nucléaire dont ne nous sommes tous bien conscients des atouts cependant la construction de nouveaux réacteurs s'inscrit dans le long terme, là où les énergies renouvelables peuvent répondre à nos besoins énergétiques, dès maintenant, le gouvernement semble avoir pris la mesure de l'urgence avec ce projet de loi qui contiennent de nombreuses mesures de simplification et d'accélération des procédures, et je m'en réjouis, mais ce texte reste perfectible, et c'est pourquoi je tiens à saluer le travail accompli au Sénat par les différentes commissions impliqué, il montre l'attention de notre haute assemblée à ce que la transition énergétique menée par l'État ne se fasse pas contre les collectivités territoriales mais bien avec elle, ma collègue daphné Ract-Madoux détaillera le point de vue de notre groupe sur les avancées proposées par la commission des affaires économiques, notamment grâce à l'engagement de notre collègue rapporteur Patrick Chauvet, pour ma part j'accueille favorablement plusieurs propositions de mon collègue rapporteur Didier Mandelli faites en commission aménagement du territoire et le développement durable, je pense par exemple à la définition à la limitation de la phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale à 4 mois ou encore au référent préfectorale à l'instruction des projets d'énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique par ailleurs ces amendements visant à démultiplier les possibilités d'implantation du photovoltaïque me semble indispensable pour maximiser le déploiement de cette énergie, cependant je déplore que certains amendements votés en commission, mettent en péril l'édifice que nous avons co-construit, comment pouvons-nous ainsi proposé de revenir sur le dispositif équilibré de la loi 3DS sur l'éolien en envisageant aujourd'hui un véto des élus municipaux sur les projets d'abord cela ralentirait la procédure, ce qui serait contre-productif. Plus dangereux encore, cela mettrait les projets éolien terrestre à la merci de critères politiques et donc subjectif, un risque d'autant plus accrues si toutes les communes en co-visibilité sont concernés aussi, je ne crois pas raisonnable ni responsable d'instaurer un tel dispositif de même comment soutenir des mesures visant à gêner l'implantation d'éoliennes Offshore à moins de 40 kilomètres des côtes quand dans le même temps l'éolien flottant qui permet d'aller au-delà de cette distance n'est pas encore mature, c'est à se demander si nous avons tous la même conscience de la gravité du moment, en pleine crise climatique et énergétique mon groupe n'étant pas unanimes sur ces questions, la vie que j'exprime représente celui d'une partie de mes collègues, nous comptons tous néanmoins sur le débat d'aujourd'hui et des jours à l'avenir pour que le gouvernement et le sénat s'accordent sur des solutions de compromis satisfaisante, je vous remercie. La parole La parole est maintenant à Monsieur Daniel Gremillet pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président. Madame la ministre Madame messieurs les rapporteurs, madame la présidente, messieurs, le président des 2 commissions, mes chers collègues. Nous avons un texte. Qui nous arrive presque un peu en urgence. Et ce texte en urgence, je voudrais en quelques. Parole retracer son histoire. Tous ont commencé avec le général de Gaulle. Lorsqu'il a fait le choix du nucléaire et de la construction de l'hydroélectricité. Tout a été poursuivi par les présidents qui se sont succédé, que ça soit le président Pompidou, Giscard d'Estaing même président Mitterrand qui, pendant un temps avait hésité, était revenu sur effectivement la nécessité de faire continuer les investissements dans le nucléaire poursuivi sous présidence Chirac. Qu'on poursuit, sous la présidence Sarkozy. Pourquoi j'évoque cela. C'est que, sans le savoir. La France était le 1er pays à avoir une énergie décarbonée pour 85 % dès l'origine, dès le départ avec le choix du nucléaire 75 % 13 % sur l'hydroélectricité. Je le dis parce que. C'est ça la réalité. Et la réalité c'est elle va encore plus loin. C'est que cette réalité, c'est aussi une réalité qui a permis aux Français d'avoir une énergie abondante et compétitif pour notre économie, à travers tous les territoires. Et effectivement. Les problèmes et les non-décisions ont commencé d'abord avec la présidence Hollande la présidence Macron. Qui, sous ces deux non mais c'est la réalité des faits parfois c'est gênant de l'entende. Et la réalité c'est quoi, on a décidé de revenir parc nucléaire. à 50 % au lieu des 75 on a décidé, effectivement, fermeture de castors serait acteur et dans les quatorze, il y avait les deux de Fessenheim où on avait dit on fermera Fessenheim quand Flamanville sera en capacité de produire. Je continue parce que. Non, ça, non seulement d'avoir décidé cela, on a aussi décidé de. Revenir sur. Astride, qui était la 4ème génération sur les productions nucléaire. Et pendant ce temps là. ça me fait penser un peu à la cigale et la fourmi. Parce que non satisfait d'avoir fait cela. Nous avons décidé d'arrêter la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur notre territoire, nous avons décidé. Le tout électrique. Et nous avons décidé aussi l'interdiction de la fragmentation, l'axe de gaz de schiste, alors que d'autres pays font ces choix-là. Le problème de tout ça, d'où ce texte d'aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas eu le en même temps il y a pas eu en même temps parce que, lorsqu'on décide de diminuer la production énergétique qui nous amène dans cette précarité que nous connaissions dans qui nous amène à ses coûts de l'énergie aussi élevés, bien plus élevé que l'Allemagne, nous sommes à 100 euros de plus que l'Allemagne, c'est du jamais vu. Eh bien, effectivement, il y a pas eu en même temps parce que on n'a pas été en capacité de produire d'autres énergies, y compris renouvelables. Et Madame la Ministre. Dans votre déclaration aux Échos d'hier, j'ai bien entendu votre propos et je voudrais vous dire tout simplement le débat que nous avons à cet instant. Quand je vois les difficultés que nous avons eu. Ici. à voter un texte notamment sur le texte climat résilience en qui disait tout simplement on ne fermera plus de réacteurs si on n'a pas l'équivalent en dur de production énergétique, c'est : on a eu des difficultés incroyable et je voudrais dire tout simplement que tous les travaux du Sénat. Qui ont été votées, ici c'est pas faute de l'voulu l'avoir dit, les travaux de la commission des affaires économiques, qui était de placer en permanence. De revenir, de garantir la souveraineté énergétique de notre pays, accessible à nos concitoyens compétitive pour notre économie, c'est des tas de propositions de textes qui ont été votées par le Sénat sur lesquels on ne l'avait pas entendu notre discours et nos propositions, donc aujourd'hui c'est un peu une séance de rattrapage, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en dehors des capacités de produire cette énergie nucléaire Nouvel horizon dans 10 ans il y a urgence à intervenir pour garantir cette énergie à nos concitoyens, merci. merci, cher collègue. La parole est maintenant monsieur Franck Montaugé pour le groupe socialiste, pour 4 minutes. Monsieur Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous l'avons dit lors d'un récent débat avec le gouvernement SMBC TPE aurait dû constituer le point d'entrée de la politique énergétique de la France au lieu de quoi nous discutons aujourd'hui sans connaître vos objectifs précis du déploiement de certaines énergies renouvelables de même du nouveau nucléaire et après-demain, peut être de l'hydraulique dans ce contexte flou et pour le moins problématique rarement un projet de loi gouvernemental aura été autant modifié sur le fond par les commissions du Sénat et leur rapporteur, que je salue et suite aux nombreuses observations du Conseil d'État et il fallait qu'il le soit, tant qu'il nous est apparu comme approximatif et imprécis sur bien des points et de surcroît de surcroît contrevenant aux libertés les plus fondamentales et des élus locaux dans la perspective d'intérêt général du zéro carbone en 2050 les sénateurs du groupe socialiste, se sont placés du point de vue des élus locaux pour améliorer votre proposition je voudrais ici rappeler notre opposition ferme à votre proposition d'ingérence des préfets dans les orientations des PLU, la solution est ailleurs, dans le respect et le dialogue avec les élus locaux pour faire avancer efficacement la production d'énergie renouvelable sur nos territoires, hein, il faut définir et déployer une planification dans le sens, État, collectivités territoriales et dans le sens, collectivités territoriales, État, nous avons dans la législation, tous les outils pour y parvenir, contrat de plan État-Région sera être Scott PCAET et PLU, j'ajoute que, bon sens et dialogue à tous les échelons, nous permettront d'être au rendez-vous des objectifs fixés sur tous les territoires, et dans les délais pour ce qui est du développement de l'éolien, nous vous ferons des propositions réalistes imprégné du vécu de terrain et de nature à diminuer l'impact des nuisances, par contre, nous pensons que le partage de la valeur doit s'opérer par l'intermédiaire des collectivités locales concernées, nous tenons à ce que le principe de péréquation tarifaire perdure pour tous les consommateurs et sur l'ensemble du territoire national, loi de Kirchhof oblige, la consommation ne se fait pas obligatoirement à proximité immédiate du lieu de production, nous tenons aussi à vous rappeler la nécessité de restructurer le marché européen et les tarifs de l'électricité. Nous tenons aussi à vous rappeler dans ce cadre, pardon, les tarifs régulés doivent être maintenus et développés, le texte permet l'accès, les collectivités locales aux contrats de long terme, type PPA, ils doivent être encadrés afin d'être protecteur, à l'inverse de ce que subissent nombre de collectivités locales, dans le contexte énergétique actuelle je voudrais aussi rappeler que mon groupe est réservé sur le nombre de critères à retenir pour qualifier l'agrivoltaïsme parmi les 4 critères proposés un seul nous paraît insuffisant, il y a un risque certain de dérive vers l'énergie culture alors que la préservation des Terres nourricières doit primer sur toute autre considération, ayant conscience que derrière ce sujet, c'est notre modèle agricole qui est en question, tout en affirmant que les agriculteurs, comme tous les Français peuvent être des contributeurs du mix énergétique nationale, c'est pourquoi nous vous présenterons un amendement visant à déployer des programmes de contrôle des installations photovoltaïques sur Culture pour terminer nous souhaiterions savoir comment les communes vont devoir prendre en compte, Lausanne dans les projets d'énergies renouvelables à cet égard, il est nécessaire d'inscrire la comptabilisation Dusan d'un jeune dispositif de solidarité ou de péréquation territoriale nationale quel est madame la Ministre votre position à ce sujet, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant Madame. Daphné Ract-Madoux pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre collègue Denise Saint-Pé s'étant prononcer sur les articles relevant de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, mon intervention ne portera que sur ce délégué au fond à la commission des affaires économiques. Je ne peux commencer qu'en félicitant notre collègue rapporteur Patrick Chauvet pour l'excellence de son travail et pour l'attention particulière qu'il a eu à essayer de trouver des solutions de synthèse, quelle que soit la technicité des sujets abordés. Les apports de notre commission des affaires économiques sont nombreux. Insertion du stockage de l'électricité dans le dispositif de la loi facilitation de la production du biogaz encouragement à la production d'hydrogène Vert ou possibilité de renforcer les capacités des installations hydroélectriques. Mais le temps qui m'est imparti ne ne permettant pas de tout traité, je me concentrerai donc sur 3 points : le 1er, sans doute le plus préoccupant pour les territoires et bien sûr l'objectif de 0 artificialisation nette le fameux Anne qui inquiète avec la transition énergétique les territoires se trouve confronté à un que l'on a un conflit d'impératifs écologiques, d'un côté, il faut limiter l'artificialisation pour préserver le milieu naturel, de l'autre, il faut construire et développer des infrastructures énergétiques pour décarboner notre mix mix est donc nécessaire d'articuler les deux pour que l'artificialisation énergétique ne phagocyte pas tout le potentiel au détriment de l'aménagement local et en l'état actuel du décret de la nomenclature Dusan il fallait impérativement sortir les infrastructures énergétiques. Très exactement ce qu'a fait notre commission sous la houlette de son rapporteur, ce faisant, elle a ouvert la boîte de Pandore, c'est le premier aménagement à l'objectif than depuis son adoption dans la loi climat et résilience. Madame la ministre, il n'y en aura d'autres, votre gouvernement s'est déclaré favorable, nous les accompagnerons attentivement avec pour ligne directrice de rendre l'objectif than applicable sur tout le territoire sans le vider de sa substance. Le 2ème point que je souhaitais aborder le partage de la valeur, un élément clé en matière d'acceptabilité des projets d'ENR, or le dispositif initial en flèche en l'intéressement sur les riverains, donner l'impression de vouloir acheter le silence on pouvait de plus crainte que ce partage ne soit dans les fêtes anecdotique, nous avons adopté en commission une réorientation qui augmente le montant du partage, puisque ce dernier est étendue à toutes les ENR et que le versement forfaitaire sera complété par une contribution territoriale Servent à financer des projets locaux de transition écologique de plus notre commission là rendu collectifs et publics, ce qui semble plus sain et logique, le dernier point que j'aborderai en conclusion est plus problématique, il s'agit de la déclinaison territoriale des objectifs de production d'énergies décarbonnées comment satisfaire nos besoins nationaux avec des projets non pas seulement acceptée mais même voulu par les territoires concernant les éoliennes terrestres, la problématique est caricatural et clivante mais elle se présente en réalité pour toutes les énergies bas carbone des centrales jusqu'au pathos panneaux panneaux pardon photovoltaïque en passant par la production de biogaz. Nous devons trouver un système de gouvernance de la transition énergétique qui conserve toujours cet équilibre entre objectifs de production et soutient territoriale, or ce dispositif, nous ne sommes loin de la voir notre commission a néanmoins commencé à poser les jalons en permettant aux collectivités qui le souhaitent d'améliorer leur planification énergétique via le schéma de cohérence territoriale le Scott et de manière simplifiée demain la programmation pluriannuelle de l'énergie devrait nous apporter un cadre global c'est, du moins telle cadre que nous appelons de nos voeux et Madame la Ministre, nous serons à vos côtés pour l'élaborer. C'est le président, Madame la Ministre, mes chers collègues, au moment d'examiner ce projet de loi, nous sommes nombreux à nous interroger tant sur sa finalité que sur les moyens envisagés. Accélérer mais pourquoi faire, dans quel but et avec quelle visibilité. Madame la ministre, notre objectif primordial est-il de limiter drastiquement nos émissions carbone. Dans ce cas, il faut bien pointer l'incohérence d'une démarche qui consiste à isoler une thématique particulière, seule celle des seules énergies renouvelables au lieu de prendre le sujet de notre mix énergétique dans sa globalité. Certes, dans une espèce de parallélisme des formes, le gouvernement nous proposera bientôt un texte analogue concernant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Mais ce texte aurait très bien pu être intégré au débat du jour avec le mérite de considérer plus globalement les forces et faiblesses de notre production électrique. Nous ne mesurons d'ailleurs toujours pas la réalité concrète de notre politique dans le domaine du nucléaire, quelle est la stratégie du président Macron à la en la matière. Celle des années 2017, 2019 conduisant à la fermeture des réacteurs de Fessenheim est à l'arrêt du programme de recherche Astride ou bien celle des années 2020, 2022 avec les annonces successives de relance du nucléaire, sans toutefois aller jusqu'à la signature de commande à ce jour, quand le en même temps se traduit par le Stop and Go, les effets sont catastrophiques. D'autre part, notre programmation pluriannuelle de l'énergie est intenable et multiplier les objectifs plus ambitieux les uns que les autres, et si possible à un horizon très lointain n'y change rien. Comme cela a été souligné par notre rapporteur Didier Mandelli redéfinir notre PPE était un préalable à toute discussion sur les orientations à prendre pour les prochaines décennies encore une occasion ratée de mener un débat de fond et si possible des passionnés. Accélérer nécessite évidemment d'avoir une certaine visibilité du point de vue méthodologique, l'idéal serait même d'avoir une feuille de route, un itinéraire clair avant de s'engager sur une voie d'accélération. à minima, connaître la direction d'un déplacement et d'une utilité certaine pour quiconque envisage de prendre la route. Madame la Ministre, initiative du gouvernement ne coche aucune case ni visibilité ni feuille de route ni direction bien identifiés et pour tout dire, même la boussole fait défaut. Mes chers collègues, sommes-nous bien certain de vouloir accélérer dans le brouillard d'une politique publique si essentielle tant pour notre développement économique que pour notre souveraineté. D'un point de vue très personnel, tout cela me fait penser à la copie d'un mauvais élève de mathématiques que le ministère de l'éducation nationale et au passage de nous dissimulé dans laquelle on trouverait pêle-mêle et sans aucune logique un tas de théorème inapproprié censé mener à une conclusion dont on ne discerne aurait plus du tout les contours aussi dans la grande sagesse du Sénat que votre gouvernement reconnaît désormais régulièrement et souligne même tout particulièrement depuis 4 mois, les commissions saisies ont tenté de remodeler ce texte pour mieux encadrer certaines dispositions, je citerai en particulier les simplifications envisagées en matière du droit d'urbanisme que les rapporteurs ont voulu davantage laisser entre les mains des élus locaux. Et le régime de partage de la valeur prévue dans l'article dix-huit ans préférant une redistribution publique et collective à une redistribution privés et individuels suspectent de vouloir éteindre le feu des contestations avec quelques piécettes emprunté au budget de la nation, je salue donc le travail des rapporteurs qui ont réussi, malgré cette confusion des intentions et cette absence de rigueur dans l'approche méthodologique du gouvernement à produire un texte plus pragmatique et plus proche des réalités du terrain, je vous remercie. Merci, cher collègue, la discussion. Qui ont générale est Close, la parole est évidemment à madame la ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, peut-être quelques mots d'abord pour saluer les apports des différents groupes dans le l'analyse de de ce texte, ce sont des avancées qui, je pense, vont contribuer à l'objectif de production de plus d'électricité bas-carbone dans les années qui viennent, mais j'entends aussi de nombreux groupes qui évoque le sujet du véto préalables des maires, je dis préalables parce que vous l'avez compris c'est un véto qui interviendrait très en amont des projets et sans qu'on ait pu analyser l'impact économique, énergétique, environnementale paysager des projets en question, il faut le nommer telle qu'il est et donc reconnaître ce qu'il fait, c'est-à-dire bloquées potentiellement des projets je je ne crois pas que ce soit l'ambition que j'ai entendu de la part de chacun des groupes qui ont pris la parole, donc je renouvelle ma proposition rapporteur le dispositif équilibré qui concilie accélération et participation des élus qui doivent avoir le dernier mot, j'ai aussi entendu vous remonter sur le sujet du traitement des dossiers et des ressources humaines, donc je veux le redire ici, oui, l'État doit se mettre en position de mieux s'organiser pour permettre le déploiement des énergies renouvelables et c'est ce que nous avons fait, comme vous le savez, nous avons d'abord renforcé le budget, vous avez la direction générale Énergie, climat est les Dreal qui ont été renforcés de 37 ETP, 37 TP c'est historique dans le budget du ministère de la transition énergétique et écologique je rassemble les deux ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu de tels renforcements d'équipes, nous avons également envoyé une circulaire aux préfets qui les mettent en position non seulement d'animer leurs propres équipes d'aller chercher des solutions d'accompagner les élus de mettre à disposition des cartographies des élus locaux pour aller plus vite et déterminé déterminé avec eux les zones qui sont le plus propice aux énergies renouvelables, tout ça est également embarqué, nous avons bien tenu compte des retours notamment du Conseil national de la transition énergétique auquel participe un certain nombre d'associations d'associations d'élus et d'associations environnementales et d'organisations syndicales et de représentants des entreprises, cette loi ne elle nous avons également pardon je le rappeler. Signé un décret sur le contentieux qui permet d'accélérer le contentieux et il est tout frais, il date du 29 octobre et il réduit à 10 mois les périodes de contentieux au tribunal administratif à la cour administrative d'appel entraînant l'absence de décision du juge un passage automatique à l'instance supérieure, voilà des décisions très pragmatiques qui montre que nous abordons la question de la production des énergies renouvelables, de la manière la plus analytique possible qu'est-ce qui bloque les projets, comment on peut lever ces blocages comment, au fond, on peut permettre, Français de disposer d'une énergie bas-carbone en abondance et compétitive en prix et j'ai donc passé à la question qui est venu sur la question de de la stratégie, mais je crois que la stratégie, vous la connaissez, vous avez même passé 3 heures j'étais malheureusement par mon Covid, mais la première ministre a été devant vous pour répondre à toutes vos questions sur la stratégie énergétique du gouvernement c'était il y a 2 semaines, la stratégie énergétique du gouvernement, vous la connaissez parce qu'en fait elle s'étaye sur les différents scénarios de RTE, et je crois que RTE été auditionné encore hier, sauf erreur de ma part. Qui sont construits sur la base d'un travail de 2 ans qui n'existe pas dans d'autres pays européens, en tout cas, et je ne crois pas qu'il soit 6 approfondie dans des pays de l'OCDE et qui pas à pas construit une par une perspective de production énergétique sur la base du nucléaire et des énergies renouvelables en donnant des potentiels en traçant des scénarios et en traçant aussi des scénarios de réduction de la consommation puisque le sujet de la sobriété, l'efficacité énergétique, vous l'avez compris sera aussi au coeur de nos enjeux énergétiques et je veux rappeler par rapport à cette boussole qui existe, qui est connu, que nous avons aussi respecter la décision du Parlement, qui veut que nous lancions un débat public très large, ce que nous avons fait ce débat public, a démarré en octobre, il fait l'objet aujourd'hui de 8000 contributions en moins de 2 semaines, ce qui n'est pas rien, ce qui témoigne de l'intérêt des Français pour ce débat, et donc non, nous n'allons pas forcer les choses simplement, nous avons un acquis, c'est la précédente programmation pluriannuelle de l'énergie, comme beaucoup d'entre vous l'ont signalé, nous sommes en retard sur les énergies renouvelables, donc faut-il attendre encore sur les énergies renouvelables, alors que nous savons tous que s'il y a un sujet sur lequel nous pouvons être d'accord et vous l'avez communément dit c'est qu'il faut accélérer sur ce sujet-là et, bien sûr, nous construirons ensemble la trajectoire de programmation pluriannuelle de l'énergie, il me semble important aussi de revenir sur un point sur l'énergie nucléaire à aucun moment depuis le lancement du programme électronucléaire, le nucléaire a dépassé 20 % de notre consommation d'énergie 20 je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a souvent une confusion lorsqu'on n'a pas on aborde les débats énergétique entre électricité et énergie, or l'énergie, c'est aussi la chaleur et c'est le carburant pour se déplacer et ce qui est en jeu aujourd'hui dans la transition énergétique, c'est précisément. De se passer du carburant, de se passer du gaz pour se chauffer et c'est là que nous allons avoir besoin à la fois de réduction de consommation et que nous allons avoir besoin de nucléaire et ce chiffre va peut-être vous surprendre mais depuis 2000, nous avons renforcé notre résilience énergétique, nous sommes moins dépendants de l'extérieur que nous l'étions en 2000 en 2000 nous étions dépendant pour notre consommation d'énergie à 72 % d'importation 72 %. En 2020, ce qui est encore plus proche, nous sommes dépendants à 65 %. D'importation, je dis pas que c'est formidable 65 % je signale juste que par rapport à la représentation qu'on peut s'en faire, on a réduit cette dépendance à des énergies importées et je pense qu'il est très important d'avoir ce débat et de ne pas confondre électricité Énergie parce que c'est probablement un des sujets qui crée de la confusion et notamment chez les Français, et donc j'appelle, moi aussi ce débat de fond des passionnés sur l'énergie, c'est celui que nous aurons en 2023 sur la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, mais vous savez déjà les grands axes de ce que nous proposerons, puisque le président de la République, il y a maintenant 8 mois, a annoncé très clairement son souhait de relancer la construction de 6 EPR nouveau, il a également annoncé son souhait de mettre à l'étude 8 EPR additionnel, il a également signifié que nous allons nous engager dans une stratégie de réduction de la consommation en se calant sur les scénarios de RTE, il a enfin précisé qu'elle était la trajet la trajectoire qu'recommandé en matière d'énergie renouvelable avec une multiplication par 10 d'ici 2050 de notre production photovoltaïque et l'installation de 40 gigawatts d'éoliennes marines tout ce débat, nous allons l'avoir il a enfin indiqué que nous prolongerons les centrales nucléaires, le au maximum, en tenant compte évidemment de la sécurité nucléaire, et dernier point sur ce sur ce sujet des centrales. Lorsque nos prédécesseurs ont lancé le programme électronucléaire, ils l'ont lancé pour 40 ans. Personne n'ignorait. Lorsque ces centrales nucléaires ont été mises en service entre 1977 et le début des années 80 que 40 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui. Nous allions passer des visites de contrôle qui allait pas durer plus de 6 mois, personne ne l'ignorez, personne n'ignore d'ailleurs que dans 10 ans, le même exercice sera fait et qu'il sera plus difficile puisque les centrales nucléaires auront dix ans de plus et comme tout équipement, il est soumis à une forme d'obsolescence lié à son utilisation et il y a une partie il y a une partie des composants qui sont remplaçables et ça on peut le faire, autant qu'on veut, il y a une partie des composants d'une centrale nucléaire qui. qui peuvent à un moment de voir ne seront pas remplaçable, c'est par exemple l'exemple de la cuve, donc tout cela est connu, sans surprise, et aujourd'hui nous devons effectivement parce que nous sommes dans une crise énergétique qui nous montre que les importations sur lequel nous avons compté depuis mai depuis le la sortie de la 2ème guerre mondiale pour prendre cette échéance là, je vais pas remonter à des temps antédiluviens ses importations, elles ne sont pas acquises, parce qu'il y a des arrière-pensées géopolitiques nous voyons avec la Russie, elles ne sont pas acquises, parce que la transition énergétique, dans lequel nous sommes engagés augmentent les prix de ses importations, elles ne sont pas acquises non plus à un prix compétitif, parce que nous payons et c'est bien légitime, le prix de la tonne carbone du pétrole et du gaz, et que c'est tout l'enjeu, que nous avons de faire face à un sujet de dérèglement climatique, donc je crois que, aujourd'hui, plus personne ne peut minorer l'impact, je vous remercie.

Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi sur les énergies renouvelables, était nécessaire dans le contexte actuel de la crise énergétique du dossier EDF qui reste à solutionner et de son corollaire, le renouvellement des concessions des barrages et des investissements à venir, mais quelle est l'ambition du gouvernement pour les énergies renouvelables, quelles sont les perspectives dressées pour le secteur, je constate une nouvelle fois que l'examen parlementaire de ce projet de loi au Sénat par les différentes commissions aura permis d'améliorer le texte et de lui donner une cohérence, en effet, il était particulièrement surprenant pour un texte sur les énergies renouvelables, de ne pas contenir des dispositions relatives à l'hydroélectricité, dont je rappelle brièvement qu'il s'agit de la 2ème, source de production électrique derrière le nucléaire avec 14 % de la production d'électricité qu'avec 49 % de la production brute d'électricité renouvelable, il s'agit de la première source d'électricité renouvelable qu'avec environ 2300 installations hydroélectriques de taille et de puissance très diverses, la France est le 2ème pays de l'Union européenne en puissance hydraulique installée pour un total de 25 5 gigawatts et 14 gigawatts totalement flexible, enfin, que la filière industrielle française de l'hydroélectricité est une filière d'excellence au rayonnement mondial composé à la fois de grands groupes et de PME performantes et créatrices d'emplois l'hydroélectricité et tu qui est une énergie renouvelable flexible et non intermittente est essentiel dans le mix énergétique actuelle, elle avait donc toute sa place dans ce projet de loi, c'est pourquoi le dépôt et l'adoption de l'amendement sur l'hydroélectricité facilitant les procédures administratives et le. est une bonne chose et je m'en félicite, merci. Merci d'avoir improvisé, la conclusion, la parole est maintenant à notre collègue Olivier Paccaud. Merci monsieur le président, élu d'un département l'Oise ou une forte partie du territoire et couverte de véritables forêts ou Bosquet éolien je souhaitais m'exprimer sur un aspect parfois négligé même oublié seule Laurence Garnier l'a évoqué tout à l'heure, celui du déséquilibre de la cartographie et de l'implantation des éoliennes sur les enseignements aussi qu'il faut en tirer, car on ne part pas d'une feuille blanche, on ne part pas d'une feuille blanche, ses profondes disparités en disent beaucoup sur les méthodes de puissants promoteurs se parent de l'habit écologistes pour accumuler de l'argent sur le dos des collectivités les plus modestes, car ce sont souvent les élus des territoires les moins favorisés économiquement qui se trouvent trop souvent contraint de céder à une forme de chantage financier n'ayant que peu ou pas de ressources, ils acceptent cette manne pour tenter d'entretenir et d'améliorer les services équipements offerts à leurs administrés, chacun pourra constater, cartes à l'appui, que les territoires les plus pauvres sont aussi les plus saturées d'éoliennes, c'est là où les entreprises ont péri que les éoliennes ont fleuri ce texte traduit d'ailleurs en son article dix-huit cette volonté d'acheter l'acceptabilité sociale et politique des projets cette générosité hypocrite nourri le mépris à l'écart de citoyens ruraux jugé réfractaire au progrès Victor Hugo l'écrivait déjà en 1869 c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches personne ni dans cette assemblée, ni dans les conseils municipaux ne s'opposent aux énergies renouvelables, mais rien ne pourra s'accomplir au détriment de la démocratie locale et de l'adhésion populaire la bonne conscience environnementale de certains ne peut faire l'impasse ni sur la qualité des Cadre de vie, ni sur la volonté des autres, lutter contre le péril climatique et environnemental, ce n'est pas non plus satisfaire les lubies de citadins favoriser qui ne subiront jamais les nuisances dues diktats éolien c'est encore moins cédé aux résolutions technocratique d'un État aveugle aux réalités locales alors, mes chers collègues, saisissons l'opportunité de ce texte pour changer la donne en redonnant le pouvoir aux territoires. Merci. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Cristina. Merci monsieur le président. L'article 1er a introduit en commission, prévoit l'introduction d'une planification ascendante à l'initiative des territoires pour le choix des sites de production d'énergie renouvelable, si je comprends bien les contraintes qui s'imposent au gouvernement son objectif, je déplore que ce texte si peu compte de l'avis de nos territoires, ces territoires dont nous sommes au sénat les gardiens, ceci nous oblige la concertation et l'acceptabilité invoqué dans l'exposé des motifs de ce texte de manière louable certainement reste ici, je le crains déshabillage verbaux : pourrait-on m'expliquer comment concertation et acceptabilité seraient améliorées avec des enquêtes publiques dématérialisée au pas de course et sans tenir compte de l'avis des populations et des élus avec des voies de recours toujours plus restreinte de même comment les éoliennes peuvent-elles devenir des atouts et des facteurs d'attractivité pour les territoires, je vous cite, Madame la Ministre, alors même qu'elles amènent la ruine touristique et la dépréciation inestimable de la qualité de vie et du foncier des habitants. Dans une démocratie digne de ce nom, qui part des territoires, la vie des populations locales doit être souverain en actes, pas juste en paroles, ce doit être, elle qui décide du devenir de leur cadre de vie et de la préservation de leur Patrimoine environnemental

conformément à notre droit un dédommagement à juste valeur avec l'encadrement juridique prévue sans inventé ce concept de valeurs partagées avec pour toute générosité la poignée, la poignée chic de la ristourne sur consommation future payé par le contribuable, alors une une accélération des et une oui mais de toutes les ENR celle montante des initiatives locales avec des projets résiliant des territoires en accord avec les populations et qui repose sur une intégration complète et objective de la décarbonation réel des projets et des coûts imposés à la collectivité, dans ces conditions, je serai très vigilante au respect de la concertation avec les habitants et les élus des territoires concernés au 1er rang desquels le maire et son conseil municipal très bien formés. Allez à la appeler terminer Madame Buffet mais je vous remercie, la parole est à monsieur. Stéphane Demilly. Le monsieur le président, la la crise énergétique que nous traversons aujourd'hui est sans précédent, restriction de gaz centrales nucléaires à l'arrêt barrage en manque d'eau après les sécheresses estivales, bref tout le parc de production électrique français sous pression et nos concitoyens sont confrontés à des difficultés inédites, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui a pour ambition de favoriser le développement des énergies renouvelables, si bien sûr nécessaire et le contexte géopolitique a fini par convaincre les plus récalcitrants, le Conseil d'État a approuvé ce texte tout en relevant que son étude d'impact était je cite insuffisante sur plusieurs articles voire inexistantes sur certaines dispositions pourtant importantes, or l'impact de ce texte peut être très conséquent pour nos concitoyens, il prévoit notamment d'alléger les exigences environnementales imposées pour installer éoliennes et panneaux en nombre et de dédommager certains riverains s'ils acceptent près de chez eux, ces sources d'énergies dites vertes, si je comprend une fois de plus, l'intérêt d'aller vite et donc la nécessité d'alléger les procédures, je souhaite néanmoins qu'on évacue pas d'un revers de main la vie des populations concernées par certaines installations, et en particulier dans ma région pour l'installation de Mazzéo lire sur ce point, je salue les avancées faites en commission, je plaide depuis très longtemps en faveur d'un droit de véto des conseils municipaux de la commune d'implantation des projets, un droit de véto, clair, pas d'une certaine manière, comme vous l'avez dit madame la ministre, lors de votre intervention dans la discussion générale car mal nommer les choses, ajoute au malheur du monde ce n'est pas une lubie que de reparler des éoliennes sur ce texte, madame la Ministre les Les Hauts de France sur la première région en terme de nombre de ma avec 28 % de puissance installée 30 % de production nationale et à certains endroits, nous sommes confrontés à un véritable mitage du territoire favoriser l'acceptabilité de tels projets ne passera pas uniquement par la distribution d'un simple chèque mais par une consultation et un accord des représentants des populations locales, on ne peut pas mettre sous couvert de l'urgence, un déni de démocratie locale, d'ailleurs, nous savons tous ici qu'une transition écologique résilientes et souveraine ne peut se faire contre les populations, je souhaite donc que la stratégie, les choix d'investissement soit élaboré en transparence, en concertation, mais elle territoire que les que les débats parlementaires qui s'ouvre aujourd'hui mère soit particulièrement constructif. on est tous d'accord, il faut accélérer et accélérer très fortement l'installation et le développement des énergies renouvelables, j'ai rien, la question n'est n'est plus là après, c'est comment on le fait et je pense que moi, je voulais d'abord saluer le travail qui a été fait sur l'article notamment sur l'article 1 à par la par la Commission sur cette nécessité sur ces mesures visant à renforcer la planification territoriale et améliorer la concertation parce que tout ce que j'ai entendu précédemment, je pense que justement on a besoin de cette planification, on a besoin de de rotation nationale et ensuite

moi je souhaitais j'avais déposé un amendement pour aller un petit peu plus loin et notamment sur le, sur la question du du solaire mais bon l'article quarante et je note d'ailleurs au passage qu'on peut même plus confier de missions sans date butoir donc Etalab dans le temps aux agents publics, des gens en poste, on peut dire que notre marge de manoeuvre devient très, très très, très étroite sur nos possibilités d'amender, mais je voulais aborder la question du concept de cadastre solaire, il me semble que, s'agissant du solaire, il faut qu'on identifie toutes les zones et notamment toutes les zones de toiture Solar Isabelle de France et qui pourrait venir justement enrichir cette cette planification il y a une très bonne échelle qui est celle des EPCI des métropoles via leur leur syndicat d'énergie et la métropole de Lyon par exemple, a fait ce travail qui a été publié en 2018 et qui me semble, hein, un exemple à suivre pour tout le monde et qui permet justement derrière de pouvoir boosté l'implantation des des énergies solaires, donc voilà, là, pour moi, la manière la plus efficace de concilier à la fois le développement des ENR et la lutte conte l'artificialisation des sols merci. Merci président la parole est maintenant à madame Martine Filleul. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, la crise environnementale que nous voyons venir depuis des années et d'où nous commençons à peine à entrevoir les effets dévastateurs nous oblige à diversifier intensifier notre mix énergétique, notamment avec l'usage des énergies renouvelables, mais cela ne doit pas aboutir à déployer de manière anarchique des éoliennes et des panneaux solaires, dans mon département : le Nord, les projets éoliens exécuté futur sont légion, la concentration est telle qu'à certains endroits, les habitants ressentent un phénomène d'encerclement et de saturation alors entendez le la concertation avec la population n'est pas accessoire et doit être approfondie pour éviter rejet recours retard et finalement échec et j'imagine mal comment nous pourrions viser l'acceptabilité de nouveaux projets d'ENR en recourant à la participation électronique et de en supprimant les enquêtes, des enquêtes publiques, le commissaire enquêteur, l'ensemble des acteurs associatifs connaissent le rôle social indispensable des commissaires enquêteurs lors de la conduite d'enquêtes publiques, il aide les populations consultées en leur rendant accessible le dossier du projet en les accompagnant, en les aidant à formuler des réponses je pense également aux phénomènes d'illectronisme qui touche 14 millions de Français, et contrairement aux idées reçues, ne touche pas que les plus âgés d'entre nous, au delà, c'est près d'un Français sur 2 qui est en difficulté avec le numérique, dès lors, la participation électronique exclut de fait une grande part de notre population, c'est dans ce sens, pour des raisons qui touche à la fois l'illectronisme et au rôle social fondamental dans dans notre démocratie environnementale du commissaire enquêteur que son intervention doit être garantie. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, renforcer la planification territoriale améliorer la concertation : favoriser la participation des collectivités territoriales à l'implantation des énergies renouvelables, nécessite la prise en compte de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, en effet, une inégalité en termes d'implantation est criante comme une saturation qui devient insupportable par endroits et le mépris des projets et des avis des élus locaux mais pris ainsi par exemple, 13 départements dans la Somme sont partie prenant de l'association Paysages et je cite de mémoire qui a l'objectif de classer au Patrimoine de l'UNESCO, les sites mémoriels du front ouest de la première guerre mondiale, l'aboutissement est conditionné à répondre aux recommandations de l'ICOM hausse de garantir un plan de gestion des sites dont celui de préserver l'environnement de ceux-ci, mais ils sont confrontés à l'obstination gouvernementale de passer outre l'avis des élus locaux qui s'oppose à ces créations, je vous renvoie au projet autour du site du Mémorial australien John Monash à Villers-Bretonneux la Ministre de l'époque, ayant refusé d'attaquer la décision de la cour d'appel, désavouant la décision préfectorale, inégalités, en outre, je rappellerai que la somme compter en juillet 2022 747 aérogénérateurs régénérateur en production 212 sont autorisés et 100 78 ans produit en instruction soit une consommation aujourd'hui de 180 hectares si nous sommes convaincus de la nécessité du développement des énergies renouvelables dans le cas du mix énergétique indispensable à satisfaire nos besoins et à garantir notre souveraineté en ce domaine, l'effort doit être territorialement et techniquement équitablement répartis ainsi le Strada devrait définir dans la concertation avec l'état et les élus locaux, les objectifs territoriaux de production des ENR avec un mix selon les potentialités locales crée ensuite une zone de développement des ENR intégré dans les épais lui auquel n'échapperait pas les métropoles et dans lequel le règlement déterminerait les objectifs, les règles de construction l'avis conforme des mers serait respectée avec la contrepartie pour la conférence des maires de s'organiser pour satisfaire aux objectifs pour atteindre ces objectifs, via les PC à ET et une péréquation fiscale qui serait délibérer ensemble décrété développer les ENR dans les éoliennes terrestres est une chose, l'organiser en est une autre et peut aboutir efficacement avec l'implication de la concertation et de l'équité territoriale si vous soutenez ces. La parole maintenant notre collègue Angèle Préville. Merci monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, oui nous sommes en retard sous les objectifs de développement des énergies renouvelables, d'autant plus que nous avions déjà et ce depuis très longtemps, pour 100 de production d'électricité grâce à l'énergie hydraulique pour les projets d'énergies renouvelables, se pose la question de l'acceptabilité d'autant plus que jusqu'à présent son développement s'est fait de façon désordonnée, pour ne pas dire anarchique et particulièrement dans mon département, c'est le cas en ce moment avec développement de parcs photovoltaïques main projets ont connu et vont connaître des leviers de bouclier non seulement la concertation est absolument nécessaire, mais doit être respectueuse de ce que sont les citoyens et des collègues ont mentionné la problématique de l'illectronisme, dont il faut tenir compte, mais également, ne faut-il pas associer davantage encore les collectivités et les citoyens sur ces projets-là et y compris financièrement, si l'énoncé du problème est très clair : il nous faut accroître la production, il nous faut aussi mesurer le changement de paradigme que constitue la production d'électricité des par, énergies renouvelables, petit rappel de physique lorsque le courant circule dans un conducteur, celui-ci s'échauffe toujours, c'est-à-dire qu'il y a perte d'une part de l'énergie sous forme de chaleur, ce qu'on appelle l'effet Joule pour limiter cette perte, un des moyens et d'élever la tension électrique, c'est-à-dire de passer sous haute tension lorsqu'on produit électricité dans une centrale nucléaire, la production d'électricité et massive, c'est-à-dire en très grande quantité on installe donc à la sortie un processus pour monter la tension, on peut ensuite distribué cette électricité en minorant les pertes par contre à la sortie d'un parc photovoltaïque ou éolien, la production est limitée, elle va être diffus sur le territoire, il est impossible de monter la tension et d'avoir des lignes à haute tension, au sortir de ces parcs, il serait donc beaucoup plus vertueux de consommer cette électricité en proximité sur place et donc de favoriser très nettement l'autoconsommation merci. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes plongés dans une crise durable, vous avez raison madame la ministre, avec des éléments conjoncturels que tout le monde a rappelé la guerre en Ukraine, le stress hydrique, la moitié de notre parc nucléaire à l'arrêt et puis des effets structurels, la libéralisation du marché, le marché européen, le fait de lier le prix du gaz à l'électricité, et je vois que beaucoup nous rejoignent sur cette question et il y a un défi d'avenir, il faudra sortir des énergies fossiles, ça va demander des milliards, des dizaines de milliards d'investissements, on a donc besoin d'un débat global une vision globale et vous, vous nous proposez de saucissonner les problèmes, on va voir ici d'abord un débat sur les énergies renouvelables, vous avez présenté hier un projet sur le nucléaire, puis viendra la PPE, mais on a un problème, on n'a pas un débat sur quel mix électrique est-ce que c'est le public ou c'est le privé qui va avoir la main et on a des manques et on a besoin d'une vision globale et je vous le dis, ce que nous allons voter là maintenant sur les énergies renouvelables, potentiellement, nous serons obligés de revenir sur la PPE, voire de se contredire et puis pour finir, nous avons 3 manque dans ce texte le 1er c'est l'hydroélectricité 11 % de notre mix électrique la plus puissante des énergies renouvelables et nous n'en parlons pas dans un grand projet de loi sur l'énergie renouvelable, la deuxième personne ne parle de ça, mais une fois que nous votons sur les ENR, avec quelle filières industrielles, nous n'en avons pas mais nous avons bien une société sur les panneaux photovoltaïques à Grenoble Photowatt qui aujourd'hui manque d'investissement même EDF qui est c'est une filiale préfère aller acheter des panneaux chinois, il nous faut ce débat et puis le dernier je vous le fini c'est sûr EDF le plus grand acteur une autre puissant outil industriel, EDF, là non plus, nous n'aurons pas le débat, puisque vous ne voulez pas et vous l'avez fait par amendement par le PLFR et pourtant je pense qu'il nous faut un vrai débat sur : quel avenir pour EDF dans les temps, Monsieur le Président remarquables. Dieu merci, merci, cher collègue là. Parole est maintenant monsieur Jean Marc Boyer. Merci Monsieur le Président, je partage et je soutiens les propos de mon collègue Olivier Paccaud tout à l'heure qui fait le constat et qui a dénoncé cette hypocrisie ambiante qui règne actuellement entre les porteurs de projets, l'administration sur l'ensemble des contraintes et des projets éoliens qui peut terrestre qui peuvent exister sur notre territoire, je veux juste donner 2 exemples est il normal aujourd'hui que une commune, un conseil municipal, un maire qui a pris position contre un projet de développement éolien de champs éolien prend position contre le préfet passe outre et accepte le projet est aujourd'hui le maire et le conseil municipal sont au tribunal pour effectivement la l'arrêté du préfet, je pense qu'il faut qu'on arrête ce genre de situation qui crée des des climats absolument délétère dans sur nos territoires 2ème exemple été le raisonnable aujourd'hui qu'un Champ éolien de 45 éoliennes en limite d'un parc naturel régional à proximité d'un site classé UNESCO aujourd'hui puisse continuer à se développer et continuer à avoir des avis favorables, je pense qu'il faut qu'on arrête cette situation-là et cette hypocrisie pour l'arrêter, je crois qu'il y a aujourd'hui 3 3 objectifs qu'il faut essayer de se fixer, premièrement, il faut que on soit dans des situations acceptable pour non seulement les citoyens mais aussi pour les maires des communes aujourd'hui les habitants et les maires des communes ne veulent plus être violée intellectuellement administrativement psychologiquement, socialement, parce que, effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la pression qui est faite sur l'ensemble de ces acteurs ne plus mettre les maires au pied du mur et quand j'ai entendu tout à l'heure, madame la ministre est ainsi que notre rapporteur Didier Mandelli dire je cite le maire doit avoir le dernier mot, alors oui, là effectivement d'accord que le maire et le dernier mot et lorsque vous rajoutez : Madame la Ministre, et là aussi on ne peut qu'être d'accord que les collectivités sont au coeur de la planification écologique

La parole est à monsieur Frédéric Marchand. Merci. Merci monsieur le président, alors le, le constat est clair et nous le partageons, nous n'avons plus le temps de prendre le temps, le constat fait il y a quelques mois par RTE est limpide, je cite, atteint dans la neutralité carbone est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables, ce développement, nous le savons bien il passe par un développement de toutes les énergies renouvelables et notamment de l'éolien terrestre alors j'entends le procès en sorcellerie fait à l'éolien terrestre et notamment dans la région des Hauts-de-France dans laquelle j'habite aussi dans le département du Nord, où on a aussi de de l'éolien terrestre mais prenons garde mes chers collègues, à ne pas hystérisée par trop le débat, nous devons être à la hauteur des enjeux dans le cadre d'une coopération renforcée entre tous les acteurs territoriaux et nationaux, et nous savons que les mécanismes existent, ça a été rappelé par différents orateurs ne tombons pas dans ce particularisme franco-français que certains adorent mais qui interpelle, nombre de nos voisins européens qui ont fait le choix maintenant depuis quelques années du mix énergétique non loin des Hauts-de-France dans un petit pays qui s'appelle la Hollande le pays de Vermeer de Van Gogh, de Jérôme Bosch de Rembrandt, tu es bien dans ce pays, on s'accorde parfaitement avec des installations d'énergies renouvelables et d'éolien terrestre, alors oui, mes chers collègues prenons garde à ne pas trop caricaturer les choses et à mon sens, dans le sens nos concitoyens attendent, merci. Merci, cher collègue. La parole est maintenant monsieur Philippe Folliot. Oui merci monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, sans énergie, il n'y a pas de vie. Et ces questions sont au coeur de préoccupations de nombres de nos concitoyens, surtout dans le contexte géostratégique que nous connaissons. J'ai en mémoire des des échanges que nous avions eu à l'Assemblée nationale, il y a quelques années, suite au Grenelle de l'environnement et du reste, où l'objectif très louable des 3 fois 20 réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, faire de telle sorte que nous puissions réduire de 20 % notre consommation d'énergie, avoir 20 % d'énergies renouvelables, forcé de constater que nous avons pas atteint cet objectif, s'il est important et essentiel de développer, je veux dire, tous les éléments de réflexion et de stratégie que nous devons avoir à la matière forcé de constater que que les choses, nous les faisons dans un ordre qui est pas un ordre logique, nous, nous, nous aurions dû avoir une grande loi relative à la programmation d'une stratégie énergétique de notre pays, comme du reste de son temps, le général de Gaulle l'avait voulu, pour notre pays et puis ensuite essayer de décliner celle-ci notamment par rapport aux éléments relatifs aux énergies renouvelables, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut développer les énergies renouvelables, la façon de se de savoir comment est de savoir si ces énergies renouvelables ce développer un lien avec les territoires avec les acteurs de nos territoires ou dans mon en fonction de directives de stratégie nationale pas accepté par les élus locaux, moi je prends un exemple dans le parc naturel régional du Haut Languedoc, il y avait un objectif qui a été atteint d'avoir 300 par exemple, éolienne, hé bien aujourd'hui on continue et on veut poursuivre aller au-delà, au mépris des positions qui sont celles des élus locaux, faut-il défigurer la montagne Noire, certainement pas, et, dans ce cadre-là, il est important de faire de telle sorte que par le biais de ce texte, nous puissions mettre un certain nombre de garde-fous pour que la parole des élus locaux, la parole des populations concernées au 1er chef puisse enfin être entendus. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Bruno Belin. Merci monsieur le président, oui : je voulais évidemment prendre la suite des des propos de notre collègue Jean-Marc Boyer il voulait qu'une François équilibré, on a bien compris qu'il fallait avancer mais effectivement regardons la carte des énergies renouvelables et, regardant la carte de France sur ce sujet là, on a oublié de citer, je l'ai pas entendu ce matin, des fois ça dépendait aussi d'estrade être donc des régions et que là aussi les collectivités peuvent être aussi s'opposer sur ce sujet-là, hé bien des communes bien des départements, on a à redire des des débats qu'ils ont avec la région, alors Madame la Ministre, vous avez dit, c'était votre dernière phrase il faut que les élus et le dernier mot, moi je voudrais que les élus et le 1er mot alors il va y avoir un débat sur l'histoire du droit de véto, peut-être que l'expression est malheureuse, peut-être qu'elle nous renvoie un ancien régime et donc que le droit de véto et et pas le la formule la mieux appropriée, mais en tout cas, il faut absolument que les maires soient ceux qui sont entendus et respectés et là, ça va nous ramener sur un autre débat et j'interviendrai dans les deux jours ceux qui vont suivre, sur le sujet, la question des ABF, je suis désolée,

Merci, cher collègue. Je ne vois plus de demandes de parole donc les prises de parole sur l'article 1 ah sont closes, en accord avec la Commission et le gouvernement, je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 14 heures 30 pour la suite de l'examen de ce texte, à savoir l'amendement 582 en 1er, la séance est suspendue.